La séance est reprise nous reprenons la discussion du projet de loi de financement. Rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 dont le Sénat est saisi. En application de l'article 47 tirer un alinéa 2 de la Constitution. Je vous rappelle que notre discussion générale est Close et que nous passons à la discussion du texte transmis au Sénat. Je crois que je suis saisie de rappels au règlement.

le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Monsieur le Ministre, ma collègue Céline Brulin, vous a demandé hier de transmettre au Sénat la vie où les votes du Conseil d'État ou les deux sur ce projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, qui peut nier ici que de nombreuses interrogations sont soulevées concernant la constitutionnalité de ce projet de loi. Selon de nombreux articles de presse, le Conseil d'État a formulé des doutes sur la constitutionnalité de certaines mesures comprises dans votre projet de loi s'est-il exprimé sur le véhicule législatif lui- même traditionnellement les avis n'était pas rendu public. Toutefois, en application d'une décision orale du président de la République François Hollande annoncé lors de la cérémonie des voeux aux corps constitués. Le 20 janvier 2015. Les avis sont sur les projets de loi depuis le 19 mars de cette même année intégralement. Intégralement rendue publique par le gouvernement sur le site Légifrance dès que les projets de loi ont été délibéré en conseil des ministres. Nous savons, Monsieur le Ministre, que cette pratique ne s'appliquait pas jusqu'à présent sur les avis sur les projets de loi finances et projets de loi de la sécurité sociale de ratification d'une ordonnance ou sur les projets de loi relatif à une convention internationale. Cette nuance révèle donc de la pratique il n'y a aucune base légale constitutionnelle a empêché le Parlement, le Sénat avoir connaissance des travaux du Conseil d'État sur le présent texte donc Monsieur le Ministre, d'une part au delà de certaines pratiques. Rien ne s'oppose à une publication des avis au vote du Conseil d'État sur peut se PLFSSR et d'autre part un doute subsiste sur le véhicule législatif lui-même ce texte aurait pu et dû relever d'une loi ordinaire. La jurisprudence Hollande si je puis dire ça. Bien Bien chacun veillera à respecter son temps s'il vous plaît 2ème rappels au règlement. Monsieur là. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce rappel au règlement, se fonde sur l'article 36 et plus fondant fondamentalement encore sur l'article 24. De notre constitution. Monsieur le Ministre, vous devez accepter notre demande de publication de la vie et des votes sur le projet de loi retraites des remarques importantes des réserves, voire des oppositions ont été formulées par la plus haute autorité de la justice administrative, la presse en effet d'ailleurs l'écho après la situation révélé par l'initiative du député Jérôme Guedj. Depuis 2015, ces avis sont publiés par convention après une décision du président de la République. L'exclusion jusqu'à présent de certains des textes comme les projets de loi de financement de la Sécurité sociale n'a aucune base Textuel. Elle peut donc être annulée d'une minute à l'autre du reste un grand quotidien du soir. Ah je le cite, révélé dans un de ses articles. Dans une note restée confidentielle. Je cite le journal jusqu'à présent l'institution du Palais Royal a suggéré de retirer certaines dispositions dont celle sur l'indice seniors que leur présence dans un texte à caractère financier est sujette à caution. Sur le plan de la constitutionnalité. L'Arctique, explique même que le gouvernement n'a pas tenu compte des remarques et a présenté le texte tel quel, mais c'est un comble. À tout de même prévu pour les articles concernés des articles législatif plus sûr pour l'avenir. c'est irrespectueux et nous vous demandons une nouvelle fois de publier ces documents. Merci de votre attention. Donner la parole à Madame Céline Bruna je note que c'était sur le même thème, le rappel au règlement de monsieur Lahellec. Madame brûle Merci monsieur le président. Mon rappel au règlement, se fonde sur l'article 36 de notre règlement et l'article 24 de la Constitution. Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas démarrer l'examen du texte sans que l'avis du Conseil d'État soit rendus publique depuis 24h nous évoquons beaucoup ici. La qualité des débats qui j'en suis convaincu. Ne se démentiront pas. Au Sénat. Mais pour que ces débats soient de qualité pour qu'il se fonde sur l'entièreté de la connaissance des éléments en jeu. Il nous faut évidemment. Cet avis ou c'est votes du Conseil d'État. D'autant que celui-ci, d'après les éléments les mots qui circulent, autant dans la presse que parce que effectivement un député, il a eu accès. Le Conseil d'État aurait émis des doutes sur la constitutionnalité de ce texte après que le président du Conseil constitutionnel lui lui-même aurait aussi émis des doutes sur la constitutionnalité d'un certain nombre d'articles de ce texte, je crois que d'ores et déjà beaucoup de doutes sont. Existe sur la procédure qui entoure l'examen de ce texte. Beaucoup de d'inexactitudes approximations voire de mensonges ont déjà été développés et je crois qu'il serait sain. Pour la démocratie et pour un examen serein de ce texte que nous ayons en effet accès au à la vie et qu'ils soient rendus publics, j'insiste parce que les parlementaires que nous sommes doivent pouvoir en avoir connaissance, mais je pense que l'ensemble du peuple français doit aussi avoir à sa cause naissance ces éléments-là. Merci. Monsieur le Ministre, vous vouliez éclairer nos 3 collègues et peut-être éclairer l'ensemble de notre assemblée. je ne voudrais surtout pas. Monsieur le Président me prononcer sur les rappels au règlement et et laisser croire que je me substituerait votre autorité pour la la police de l'Assemblée de nos débats. Mais sur le fond puisque j'ai été interpellé. Peut être faire 3 remarques avant d'aller à la réponse. La première remarque mais je la fais avec le sourire. Si vous m'interrogez, toutes et tous sur un document resté secret dont vous connaissez la teneur. C'est la particularité en renvoyant parfois. en renvoyant parfois. À des brèves rapportée par un hebdomadaire satirique mais ça fait partie du du débat. La la 2ème chose pour dire qu'une partie de la réponse est dans la question que vous avez posé. Sur une décision râle. Il a été décidé en 2015 et si du président de la République de rendre publics les avis concernant les projets de loi ordinaire. Cela ne concerne pas, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, ni les projets de loi de finances, ni les projets la finance rectificatif ni les projets de loi de financement de la Sécurité sociale et il n'est pas de mon autorité de changer cette règle puisque cette règle a été fixée par le président de la République précédent et je ne me hasarderais pas de telles décisions. 3ème remarque lorsqu'il s'agit. D'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale comme d'un projet de loi de finances. Le Conseil d'État ne rend pas d'avis. Il remet au gouvernement et en l'occurrence au secrétariat général du gouvernement. Une note de synthèse. Cette note de synthèse n'est pas un avis, je le répète et les remises au secrétariat général du gouvernement. Il se trouve qu'un certain nombre de parlementaires par les fonctions qu'ils exercent peuvent s'ils le souhaitent demander à consulter cette note auprès du secrétariat général du gouvernement, dans des conditions prévues par celui-ci. Voilà la réponse que je pouvais faire. Monsieur le Président. Madame Lienemann vous voulez faire un rappel au règlement. Oui, chers collègues. Toujours au, au motif de l'article 36 de notre règlement intérieur. Madame Aubry disait historiquement quand il y a du flou. Il y a un loup. Et donc ben la gare où. bref. Vous m'avez compris, Monsieur le Ministre. Vous nous indiquer. Que le précédent. Président de la République. Refixer une règle. Je m'excuse les les du président de la République ne sont pas des lois, ce sont peut-être des us et coutumes mais ça n'a pas valeur législative qui s'impose. Heureusement nous ne sommes plus en royauté. Bon. Deuxièmement, vous, vous nous dites qu'il est possible de consulter les notes de synthèse. Mais pourquoi les cacher. Vous nous avez fait d'ailleurs vous chers collègues de l'air des grandes déclarations pour 10 explique le référendum, c'était pas bien parce qu'il fallait consolider la démocratie parlementaire. pour que le parlement délibère. Il doit être réellement éclairé par le gouvernement. Or le gouvernement lui cache manifestement des éléments qui ont été mises à en sur la table par le Conseil d'État et s'ils nous les cachent, ce n'est pas par hasard c'est que a priori il y aurait un certain nombre d'articles prévue dans cette loi qui ne sont pas conformes à notre constitution et ses articles. Même à supposer qu'ils soient pas le coeur de cible, à savoir l'allongement de la retraite avec un départ à 64 ans. Constituent le gros de votre argumentaire pour nous dire c'est pas catastrophique, on a mis des rustines, puisque par exemple, l'indice senior et cetera et cetera vous trompez donc par votre manque d'informations. La la délibération de notre assemblée, et par là même les Français. Présidente Laurence Rossignol. et se fonde sur les articles 5 et 20 de la Constitution. Monsieur le ministre Olivier Dussopt, hier vous avez déclaré au Sénat. Je vous cite, si nous sommes dans le cadre de l'Arctique 47 hein. Ce n'est pas une décision du gouvernement, l'article s'applique à l'ensemble des lois de finances et vous vouliez ainsi justifié le temps contraint de l'Assemblée nationale comme si en fin de compte, tout cela n'était pas de votre faute et cool, vous étiez totalement. Passif à l'égard de la Constitution. Or, je vous rappelle qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. La décision. 82 cas de 1986 décision 86 209 qui précise très exactement que le fait de ne pas de déférer à ses prescriptions. Et de laisser l'Assemblée nationale statuer sur un projet dont elle n'est pas dessaisi ne constitue cependant pas une irrégularité de nature à vicier la procédure. Et le constituerait une que s'il avait pour conséquence de réduire le délai dont disposent au Sénat. Si je vous la fais plus simple vous pouviez tout à fait laisser l'Assemblée nationale dans le cadre de l'article 47 hein. Continuer de débattre à condition que vous laissez au Sénat le temps. Imparti au Sénat est due au Sénat. Rien ne vous en empêcher. Dans ce cas, l'article 47 hein. Nous vous imposez pas ce que vous avez dit hier donc mon rappel au règlement vise ne sais pas la tête dans un sens de droite à gauche c'est-à-dire négativement mon interprète mon interprétation et. De gauche à droite, mes collègues me disent voilà et quand vous O'Shea tête de gauche à droite fait attention qu'elles reviennent parfois au milieu. Et donc, ce que dit mon rappel au règlement, c'est que je vous demande, monsieur le Ministre, dans la suite de ces débats de ne pas manipuler et tendre la constitution à votre seul Avantage et d'en respecter la lettre et ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Madame pour ces mange. Merci monsieur le président. C'est donc un rappel au règlement, au titre de l'article 17 bis ou 45 de notre règlement intérieur la discussion de la réforme. Commence mal. Elle est largement entravée par les centaines d'irrecevabilité. Qui frappe nos amendements. Cette loi qui traitent insuffisamment des questions de travail via un simple index senior ne peut pas être amendé en ce sens qu'a beaucoup des amendements permettant l'amélioration des conditions de travail, la prise en compte des critères de pénibilité redéfinition de certains seuils. Au coeur des questions de pénibilité d'inaptitude et donc de retraite ont été déclarées irrecevables au qui ne porterait pas sur une loi de financement de la Sécurité sociale. Mais alors c'est que si ça ne se qui ne traite pas des financement de la Sécurité sociale, c'est alors l'index senior auquel ces amendements étaient rattachés. Et cet article se trouve donc quasiment inamendable, c'est nouveau, on nous empêche aussi demander des rapports sur la décote ou de parler des caisses de retraite dans une loi réformant les retraites certains amendements ont été repris du PLFSS précédent qui n'avait pas été déclarée irrecevable comme celui de la PCH qui avait figuré dans les 3 derniers paient. Projet de loi, on nous empêche également d'aborder certains sujets sous l'Ondam alors que nous sommes sur un PLFSS, paraît-il, ou bien nous sommes face un PLFSS et dans ce cas il faut le traiter comme tel, ou bien il faut d'ores et déjà pouvoir assumer que le véhicule actuel n'est pas approprié. En tout état de cause, la mère des réformes devrait pouvoir nous faire débat des conséquences qu'elle aura sur le travail, la pénibilité, le système de soins les finances les recettes. Par contre je note que des amendements de dépenses de la droite sénatoriale sont acceptées. Ah ben ça c'est un vrai comble. Hé oui c'est pourtant cela donc c'est totalement vous commencez très mal cette discussion et nous allons en tenir compte.

Monsieur le Ministre hier après la la fin de la discussion générale, lorsque vous avez répondu aux interventions. Vous avez indiqué que le fait que le temps soit encadré ou limité n'était pas de la responsabilité du gouvernement. j'espère ne pas vous l'apprendre. Il est possible de réformer le régime des retraites sans passer par un PLFSS d'ailleurs c'est ce qui fut fait pour les lois de 2013 dites Touraine et la loi de 2010, donc c'est bien. Choix du gouvernement qui a été fait, pourquoi nous, nous en apprenons à chaque instant vous avez indiqué tout à l'heure que la particularité des Plfss était qu'il n'y avait pas d'avis du Conseil d'État. Il faut dire que ça tombe bien, d'autant que les avis du Conseil d'État effectivement sont traditionnellement publiée qu'il y avait simplement une note dont nous n'avons pas compris si bien qu'étant secrètes, vous acceptiez de la communiquer, mais j'ai l'impression, pourtant que la réponse serait non. Ensuite, nous le savons tous, vous savez, ainsi qu'avec le PLFSS, vous pourriez avoir accès aux fameux 49 3. C'est dire la confiance que vous avez dans le vote de l'Assemblée et vous avez la possibilité d'encadrer les débats et c'est là que cela vous intéresse, je rappelle que l'article 47 tirer hein. Ne vous impose pas de limiter le débat le 12 mars puisque vous pouvez le poursuivre encore pendant certains jours, sauf si votre rêve c'est de pouvoir mettre en place cette réforme des retraites par ordonnance c'est peut être finalement la volonté du gouvernement depuis le début. Donc Monsieur le Ministre, nous avons appris beaucoup de choses de votre part au fur et à mesure, nous devions avoir 2 millions de personnes bénéficiaires de la retraite à 1200 euros. Ils ne sont plus que 13.000. Qui sait. Peut être avez-vous aujourd'hui découvert que le PLFSS et le recours à cette procédure si particulière était en fait malicieuse de la part du gouvernement. Monsieur Meurant. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce sujet est un sujet compliqué comme on pourrait avoir pu le dire hein. Marc Laménie ou un sujet. Complexe comme l'a dit hier Monsieur le Ministre Dussopt. Il y a un sujet complexe. Peut dire qu'il faudrait avoir un peu de temps. Pour apprécier. Et avoir un recul sur la réforme en cours. Et les retraites, c'est un héritage. Dis à notre histoire et un héritage qui est plutôt réussi à sans reprendre une chanson de Pierre Perret. La retraite des vieux c'est plus que ça a été on a pu faire progresser. Il a éliminé la plupart des pauvres chez les anciens. Ça touche vraiment tous les Français, il suffit de voir ce qui se passe dans les rues pour s'en apercevoir, alors comment convaincre et persuader les Français sans avoir le temps. La première condition, effectivement, c'est de respecter le Parlement et l'article 47 hein à ce titre à mon avis et d'une faute. Utilisation de cette procédure pour accélérer le débat est une faute politique et c'est pas loin d'un détournement de procédure, comme le disait hier, notre collègue Kader. Faute devant le parlement mais faut tous faute devant les Français qui sont inquiets et ils sont légitimement inquiets, vu le succès et vu le peu de confiance qui font dans la parole publique politique. Des partis politiques également de ce qui se passe dans les différentes assemblées. Comment justifier sur le plan des idées, le passage d'une réforme systémique révolutionnaire de 2019 et moi je me méfie moi des conséquences des révolutions à une réforme paramétrique à certainement des éléments positifs mais dans laquelle ce qui retenu et ce qui est devenu totémique. C'est l'âge de départ en retraite.

Bien sûr que non. Et je crois que pour faire. Je conclus Monsieur le Président, qu'il faut parfois et ça va faire plaisir à, c'était parti de l'hémicycle, savoir donner du temps au temps et ce qui est certain c'est que la politique comme art de mener le changement est définitivement mais vous incompatible avec le en même temps. Dernier rappel au règlement, madame la présidente Assassi. Oui mais. J'ai été surprise. Merci Monsieur le Président je reviens c'est un rappel au règlement aussi fondé sur. L'article je sais plus lequel. Mais mais quand mes camarades blond cité tout. Hier nous avons vous nous en avait inventé hein donc c'était très bien,

Émises par mes camarades sur l'avis du Conseil d'État dont nous avons pris connaissance pour partie effectivement dans dans dans la presse. Je souhaiterais, Monsieur le Président que nous puissions avoir une suspension de séance pour permettre à Monsieur le Ministre, de téléphoner à ses services afin que ceux-ci lui fasse parvenir les documents et que nous puissions en prendre connaissance. Madame la présidente, vous vouliez répondre sur le plan téléphonique on ne suspendra pas. Je, je suis clair toute de suite madame. Un président de la commission. je la parole m'a été donné. Donc je vais la prendre. Merci monsieur le président et je vais être un peu long et je demande l'indulgence du plateau mais je pense que les interpellations sur les six recevabilité appelle une réponse détaillée. Grâce à la récente notoriété acquise par l'article 47 1 de la Constitution que nous appliquons chaque année à l'Automne pour l'examen de la loi de financement de l'année à venir. Nul n'ignore désormais que la réforme des retraites est porté par un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les règles de recevabilité des amendements pour ces 2 textes sont fixées par la loi organique du 14 mars 2022 codifié par le code de la sécurité sociale. Le règlement du Sénat me confie la lourde tâche d'appliquer ces règles et je tiens à rappeler que ce n'est un exercice plaisant qu'un président de commission qui en a la charge. Mais il s'agit d'une obligation constitutionnelle. que j'ai dû exercer cette année dans des conditions particulièrement éprouvante de délai et du nombre d'amendements. Je veux tout d'abord rappeler que les règles de recevabilité découle directement des délais constitutionnels d'examen des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, garantir la recevabilité des amendements. Une façon de s'assurer que le Sénat dans le délai qui lui est imparti délibère sur des amendements qui ont effectivement leur place dans ce texte. Il s'agit donc d'une réforme des retraites portée par un PLFSS P. L. F R SS et non d'une loi retraite née d'une loi travail 1er critère de recevabilité, il faut que les dispositions proposées à un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale comme à l'accoutumée, les amendements qui portent sur des dispositifs ne relance relevant pas de la sécurité sociale mais des régimes complémentaires de l'assurance chômage de l'État ou encore des collectivités locales ne sont pas recevables les dispositions portant sur le droit du travail sont irrecevables qu'il s'agit de la négociation collective, l'emploi des seniors CPF santé au travail même si pour l'article 2 dont le sort. Duquel soumis au Conseil constitutionnel. La présence dans le texte ne suffit pas à assurer la recevabilité des amendements portant sur ces sujets sur la cadette. Je signale que l'objectif d'amortissement de la cadets ces deux rangs organique, sauf à le remettre en cause ce qui serait recevable toute privation de recettes doit donc être comment compenser par une recette assis sur l'ensemble des revenus sur l'information des assurés. Le Conseil constitutionnel censure régulièrement des dispositions au fil des PLFSS. J'ai donc déclarée recevable ensemble des amendements qui s'y rapportait beaucoup d'amendements et j'en viens au rapport porter enfin sur des demandes de rapport au gouvernement. de la de la position défavorable de la commission de telles demandes. J'ai apprécié la recevabilité de ces amendements au regard de la jurisprudence très strict du Conseil constitutionnel qui retient lecture rigoureuse de l'article L O 111 tiret 3 12. Cet article prévoit que la loi de financement de la Sécurité sociale rectificative peuvent contenir des dispositions améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale. Et j'insiste sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, c'est-à-dire des dispositifs bien identifié des rapports prospective qui ont pour seul objectif de se conformer à l'article 40 de la Constitution et demande évaluation d'hypothétiques dispositif ne saurait relever l'application de la loi de financement de la Sécurité sociale. De même les amendements qui bien que mentionnant l'application des la FSS comme un gage de recevabilité portait en réalité sur des effets lointains diffus ne saurait être apprécié comme recevable. Ils peuvent être remplacés par des prises de parole et en le même homme Shell, même effet. J'ai ainsi examiné près de 450. Amendements portant des demandes de rapport 450 amendements, ce qui représente 9 et demi pour 100 des amendements déposés 251 ont quand même été déclarés et il a été déclarée recevable, il en reste donc près de 200 examiner ce qui représenterait potentiellement déjà beaucoup de lecture la règle son donc les mêmes quand PLFSS mais avec une contrainte supplémentaire que les amendements proposés effectivement un effet en 2023 pour ce qui est d'une loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif les recevabilité prévue à l'article L O. 111 tiret 3 12 du code à la sécurité sociale. De temps plus strictes que les faits indispensable sur les comptes des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale se doit d'être sensible l'année en cours donc tout amendement porte un dispositif prenant effet au-delà de 2023, repoussant après 2023 l'application d'un dispositif proposé a été ainsi considéré irrecevable. Voici les éléments d'explication que je sois. Apporter et je voudrais pour terminer sur l'ensemble du test, 780, 13 amendements ont été déclarés irrecevables au lieu, au titre de la loi organique relative aux lois de financement sur les 4734 déposées, soit 10,4% et un taux très légèrement inférieur à son constatés en LFSS. Il reste donc plus 3700 amendements à examiner. Et le débat aura bien lieu. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on met un rapport ou comptes sociaux que c'est recevable. Merci. Nous allons maintenant passer à une motion de renvoi partiel que a été déposée par. Madame Corinne des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain. Tendant au renvoi la commission de l'article liminaire Madame Ferré.

Le présent article liminaire entérine une réforme des retraites, commandé par l'impératif d'équilibrer les comptes publics. Suite aux nombreux cadeaux fiscaux accordés par le gouvernement aux ménages les plus riches via la suppression de l'ISF ou l'introduction de la flat tax, mais aussi aux grandes entreprises avec la suppression de la CVAE notamment ce même gouvernement cherche à nous imposer sa réforme paramétrique en usant de l'article artifice de l'article 47 tirer 1 de la Constitution et en passant par un budget rectificatif de la Sécurité sociale pour réduire à peau de chagrin. Nos travaux ce recours à une loi de financement plutôt qu'un projet de loi ordinaire, fait que les sénatrices et sénateurs n'ont pas eu l'occasion de débattre au stade de la commission et de poser véritablement la question des recettes. Cela aurait permis par exemple de se pencher sur l'excès d'exonérations de cotisations sociales dont certaines sont sans aucun effet notable sur notre économie mais coûteront à la branche vieillesse 18,9 milliards d'euros en 2023, soit un peu plus que le 17, 7 milliards que le gouvernement dit chercher d'ici 2030 à travers sa réforme avec un système de retraite qui collecte, plus de 300 milliards d'euros par an et dans un contexte où le gouvernement est capable d'augmenter les dépenses ou de baisser les prélèvements à coups de dizaines de milliards, trouver des solutions avec un objectif de justice sociale ne devrait pas être bien difficile. Revenons donc sur les baisses d'impôts injuste taxons les super profits soumettons à cotisation patronale les revenus issus des dividendes ou des rachats d'actions. L'effort ne serait acceptable que si les partagé, partagé par tous. Nous avions déjà rejeté le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Nous vous avions messieurs les Ministres notamment également alerté sur le poids de l'inflation et sur l'insuffisance du rehaussement de l'Ondam pour nos hôpitaux publics particulièrement et même aujourd'hui avec plus de 750 millions de plus, c'est insuffisant. Pour toutes ces raisons, nous vous nous considérons qu'il y a lieu de renvoyer à la commission l'article liminaire du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure générale. La vie est est défavorable. Je remercie ma collègue Corinne Ferré. D'avoir autant de de enfin de penser que la Commission pourrait encore travailler sur le sujet, je pense que nous avons suffisamment débattu et c'est une question qui concerne. Surtout. Les lois de financement de la Sécurité sociale, que nous débattons chaque année et donc ce sera. Un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre-t-elle. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs et sénatrices évidemment avis défavorable à cette motion tendant à opposer le renvoi en commission. Ce texte est évidemment absolument crucial pour que nous soyons en capacité de continuer à payer les pensions de nos retraités chaque mois. Cet article liminaire est également aussi crucial pour cela et j'ajoute qu'il est aussi crucial pour notre hôpital public. Dans cet article liminaire figurent les moyens supplémentaires que nous mettons pour l'hôpital public en 2023 à la suite des annonces du président de la République, notamment pour le revaloriser le travail de nuit. 600 millions d'euros de plus en 2023 pour l'hôpital public pour financer le travail de nuit et donc en fait en voulant renvoyer cet article liminaire en commission. Vous voulez au fond écarter ses moyens en plus pour l'hôpital public. Évidemment ça n'est pas notre objectif. Et pour ces raisons. C'est un avis défavorable. Nous allons passer aux explications de vote Madame Monge. Merci monsieur le président. Nous savons, monsieur Attal, que si on ne veut pas cette réforme les trains désormais déraille rond et en plus qu'on vaccinera pas les enfants et caetera, bon si vous pouvez nous passer tout ça. Mes chers collègues, que les choses soient dis dès à présent le groupe écologiste soutient amplement la motion présentée à nos par nos collègues socialistes, la réforme des retraites examiné répond selon le gouvernement. Un impératif d'équilibre des comptes publics, mais ça c'est à moyen terme puisqu'elle a, elle, coûte en fait 400 millions en 2023. De façon nette cette loi donc pose quand même et nous y reviendrons plus tard. De nombreuses questions sur les notamment les tableaux de financement, les méthodes de financement tout autant. Bien sûr qu'elle n'a pas que le monde du travail sans que l'on puisse en parler de façon satisfaisante, nous l'avons vu avec la suppression des amendements, c'est donc le débat doit prévaloir. Si la situation est suffisamment grave pour justifier le débat que nous avons ici, alors il faut que la discussion puisse avoir lieu sur des des bases. Discuter suffisamment et que le temps nécessaire et soient consacrés en conséquence, nous soutenons la motion. De nos collègues socialistes. Pour le groupe socialiste. Madame Pumerole, je rappelle qu'il y a une seule explication de vote par groupe hein. Merci monsieur le président. Je serai donc je serai donc la seule. Je voulais bien sûr. Confirmé la volonté que nous avons de ce dans cette demande de renvoi en commission. Vous êtes tous des élus locaux, départementaux et cetera et vous savez combien le travail en commission est important et combien il permet d'avancer dans le dossier puisque c'est en commission. Comment le général que l'on font un petit peu les principes qui seront ensuite vu au au cours de la. au cours de la session aussi lente. Dans le cas précis de ce texte. Nous avons eu des réunions de commissions qui ont consisté à dire. Avis favorable défavorable sur une série d'amendements. Ça peut nous puissions discuter ni une seconde sur le fond de ces amendements, il n'y a pas eu de discussion sur le fond, il y a eu simplement l'avis défavorable pour ne pas dire exclusivement défavorable sur tous les amendements que nous avons des pas déposer mais jamais. De discussion sur le fond. Or, discussion sur le fond et sur le fait que ce serait une réforme n'est qu'une façon effectivement de masquer le déficit des comptes publics qui sont présentées donc par. Nos 2 ministres. Je crois que il ce lieu aurait mérité vraiment d'avoir une discussion. En commission et c'est pour ça que Lucian cette. Demande. D'autres explications de vote. je vais donc. Consulter le Sénat sur la motion de renvoi de l'article liminaire, ceux qui sont favorables à la motion de renvoi. Proposée par les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain le manifeste en levant la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Et nous passons à l'article liminaire. Sur lequel je suis saisi d'une serre dit de demandes de parole tout d'abord pour le groupe communiste républicain citoyen Madame, Cathy. Ah pour ce. Merci monsieur le président. Quelles. Quelles raisons vous conduisent à faire en ce qui concerne le gouvernement et à soutenir en ce qui concerne la majorité sénatoriale, cette contre-réforme, premièrement, la mise en oeuvre des obsessions de longue date des institutions de l'Union européenne au 1er rang. Desquels la commission un règlement européen du 20 juin 2019, créer un produit panne panne paneuropéen d'épargne-retraite individuel. Le gouvernement s'est réjoui de ce nouveau produit dans dans un texte voté par le Sénat. Il y a moins d'un mois. Ce règlement, détaille le dessein européen pour tous les États membres qui tenteraient de lutter contre la capitalisation contre la privatisation de l'assurance-vieillesse alinéa 16 cette proposition jettera les bases d'un marché plus sûr, plus rentables et plus transparentes, produit d'épargne retraite facultatif d'un coût abordable pouvant être à l'échelle pas ne. ben dis donc ce projet de règlement dans une forme de déni total de la réalité des travailleuses et des travailleurs européens affirment que les limites à la portabilité des produits d'épargne retraite pose des difficultés dans l'exercice de leurs libertés fondamentales en étant par exemple empêchées d'accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État-membre, la retraite par capitalisation mais de préférence. S'il vous plaît comment sinon c'est peuvent travailleurs pourraient-ils prendre leur retraite. S'ils ne peuvent jouir de leur économie dans un autre pays. Toutes ces décisions sont déconnectés de la réalité des travailleuses et des travailleurs du pays. Un marché à 2100 milliards d'euros ici 2030, selon le cabinet de conseil d'audit, et seulement si, les avantages fiscaux suivent le projet politique est clair, faire payer aux travailleurs les baisses d'impôts aux entreprises ou injuste au ménage voyez pour 2023. merci Monsieur le Président. Mais messieurs les les ministres, mes chers collègues. On a eu un écho tout à l'heure mais c'est vrai que l'article liminaire n'est n'est pas là par hasard. Parce que liminaire, ça signifie qu'il est placé au début et pourrait être un peu plus évocateur vu le sujet qui concerne et qui forment le commencement de quelque chose qui prélude à quelque chose et on va y venir. Cet article liminaire, hé bien le point de départ, vous avez raison monsieur le ministre Atal et il est crucial. C'est le point de départ de votre réforme. Faut avoir l'honnêteté de reconnaître ça et c'est un élément de justification. C'est après que ça va coincer. C'est que le solde des administrations de la sécurité sociale est prévue en excédent de 0 eu 8 points du PIB en 2023 la dont acte. On est OK. Et moi je vais vous dire là il y a un problème de paradoxes et j'appelle ça même une étrangeté politique. Quand on sait que c'est précisément le déficit du système de retraite et se compter en 2046 dans le rapport du conseil d'orientation des retraites. Selon le scénario qui est retenu par votre gouvernement donc l'article et bien le point de départ crucial de la réforme des retraites car l'évolution de la dépense publique des administrations sociales en 2023 diminue une fois retranché l'inflation, une fois qu'on y retranche l'inflation d'un point de PIB. Ça veut dire quoi. Mes chers collègues. Un point de PIB, c'est précisément 25 milliards d'euros, 25 milliards d'euros, c'est près de fois. Le déficit du système de retraite estimait en 2046 et je vais aller plus loin parce que ayant des ambitions et plus que deux fois le déficit attendu en 2030, donc sans baisse en volume des dépenses de la Sécurité sociale si l'intégrité était reportée sur la branche vieillesse, alors nous pourrions ouais nous pourrions absorber les déficits du système des retraites et je vais vous dire, pour les années 2020 cas, 2025 2026 et je répète, si en 2023 ont dépensé en volume strictement ce qu'ont dépensé l'année précédente pour la sécurité sociale, on pourrait rayer d'un trait de plume les déficits du système des retraites en 2024, 2025 2025, dont le vote architecture financière et comptable s'écroule et c'est l'effet vous conclut oui je vais conclure j'ai posé une question, je la poserai pendant les 12 jours. Vous me direz, l'amendement de la droite attendez a terminé j'arrête. Très bien monsieur le président. Poncer Monge. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à messieurs les Ministres préalablement je voudrais un éclaircissement quant au tableau de la synthèse des mesures de votre réforme vous annoncer que votre réforme rapportera 17 7 milliards supplémentaires au régime des retraites bien les mesures paramétriques de votre forme sont bien l'accélération de la durée requise le passage de 62 à 64 sauf pour les invalides ou les inaptes qui reste à 62 ans et les personnes handicapées qui reste à 55 ans, un gain financier de 17 7 milliards. Sur ce, sur lesquels s'appliquent les mesures paramétriques. À cela vous soustrayez des mesures d'accompagnement qui génère des coûts supplémentaires. Revalorisation des Mikko validation de trimestres. Bref, des dispositions qui n'existe pas dans la loi actuelle et qui donc réduisent les gars de votre réforme. Mais vous soustrayez également le maintien le maintien, pour les personnes invalides ou inaptes à hauteur de 3,1 milliards alors que cela ne change absolument rien à la situation d'aujourd'hui ils basculait dans la retraite à 62 ans et c'est toujours le cas avec la réforme, la trajectoire du système de retraite n'est en rien modifié pour en cela sur ce plan, la réforme n'apporte ni gain ni coût différentiel. Le coût de ces pensions des 62 ans, était déjà présente dans les projections du système de retraite, avant la réforme et resteront inchangés après la réforme. Ils n'ont donc pas apparaître dans ce tableau qui ne concerne que l'impact des recettes et des coûts de votre réforme Monsieur le ministre, messieurs les Ministres, pouvez-vous m'expliquer ce qu'un maintien donc une absence de mesures ni plus néanmoins fait en fait dans un tableau de synthèse financière de l'impact des seules mesures de la réforme. Monsieur Christophe André Frassa. de minutes pour vous parler des grands oubliés de cette réforme des retraites, les Français ayant effectué une partie de leur carrière en France et à l'étranger. Les problèmes rencontrés sont de 3 ordres et concerne la garantie de la continuité des droits entre nos systèmes de retraite français et le système des autres pays. Première difficulté, certains pays n'ont pas signé de convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France. Il en résulte que les années cotisées dans ces pays ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la décote. Le montant de la retraite française peut se trouver en conséquence minoré de 25 102ème difficulté l'impossibilité de prendre en compte pour le calcul de la décote, les années cotisées dans plusieurs pays non-européens. Si vous avez effectué une partie de votre carrière en Égypte et aux États-Unis, vous devrez opter pour comptabiliser les années effectué dans l'un ou l'autre mais pas les deux. C'est une injustice qu'il convient de corriger car il en découle des inégalités selon les pays dans lesquels vous avez effectué votre carrière professionnelle, nous n'avons pas pu présenter d'amendements permettant d'échapper à la décote dans ce genre de situation, car il aurait été déclarées recevables au titre de l'article 40. À défaut, nous avions déposé un amendement prévoyant la présentation d'un bilan annuel devant l'Assemblée des Français de l'étranger. Concernant les accords de sécurité sociale avec les pays non-encore conventionnés. Cet amendement a lui aussi été déclarée recevable, nous en prenons donc acte 3ème difficulté enfin se pose la question du salaire de référence pour le calcul de la pension de retraite lorsqu'il porte sur les 25 premières années les meilleures années si la la carrière effectuée en France a été d'une durée égale ou inférieure et qu'elle concerne les premières années d'activité. Le montant du salaire de référence sera le plus souvent assez bas, là encore, il conviendrait d'étudier ces situations et d'envisager des mesures, des mesures des mesures correctrices tels qu'une proratisation du décompte ainsi une personne. À exercer je je conclus tout de suite pendant 10 ans en France, le salaire de référence pour le calcul de la retraite devrait porter sur les 6 meilleures années effectuer une partie de sa carrière professionnelle international c'est une réalité, ce n'est pas pris en compte

Merci monsieur le président. Chers collègues, Monsieur le Ministre. Cet article liminaire fond de votre réforme des retraites sur le solde budgétaire de la sécurité sociale et ce solde est exprimé en référence au seul indicateur du produit intérieur brut pour nous sanctuarisé cet indicateur est réducteur. Nous ne pouvons penser l'efficience de nos politiques publiques en la référant au seul critère quantitatif du PIB. Le PIB pour être simple et connu de tous, n'en est pas moins très incomplet et il ne dit rien sur la pénibilité du travail sur l'espérance de vie en bonne santé, pour ne citer que ces 2 aspects du sujet d'éminents économistes comme Stiglitz Sen Fitoussi, on fait une critique radicale du PIB comme instrument de mesure centrale de la richesse d'un État ou d'une nation. Non un État n'est pas riche du fait seulement de son PIB, le PIB ne rencontre que très imparfaitement de la place centrale, que la sécurité sociale occupe depuis 1945 dans notre société et dans le contrat social qui nous lie tous les uns aux autres, y compris, Monsieur le Ministre pour les bien nés, où les nantis vers qui vont en permanence les valeurs les faveurs politique de votre gouvernement une réforme juste doit être inspiré par la réalité de ce qu'il fait pour nous, société et pour cela, le gouvernement devrait prendre en compte un panel de nouveaux indicateurs de richesse d'inégalité ou de qualité de vie qui traduisent que certains que ce que certains appellent et je les salue ici le pouvoir de vivre l'indifférence de votre gouvernement à prendre en compte les difficultés de la vie réelle des Français est profondément dogmatique. Pour ces raisons, j'appelle avec mon groupe a rejeté cet article liminaire dans le référentiel était inadéquat au sujet des retraites.

la note de synthèse du Conseil d'État parce que je pense que sur tous les bancs de cet hémicycle, on doit quand même espérer que les sénateurs et l'ensemble des éléments pour débattre en toute sincérité et en toute objectivité. L'article liminaire. Cet article fait référence à une loi qui n'a pas encore été approuvé la LPFP. C'est à cette occasion que j'ai d'ailleurs entendu pour la première fois parler de l'enjeu de cette réforme des retraites par le ministre Bruno Lemaire qui citait que cette réforme était un des effets hein des efforts structurels indispensable pour rétablir le déficit public à 3%. Le caractère de réformes d'austérité de cette réforme des retraites était parfaitement assumé par le ministre Lemaire. Donc je voudrais savoir où est la loi de programmation des finances publiques car dans cette loi pas adopté. Nous avions ici même voté un amendement qu'à gauche, nous avions tous ceux qui ont battu de suppression de 120.000 postes de fonctionnaires. Je ne retrouve pas la suppression de ses 120.000 postes de fonctionnaires à l'intérieur du tableau qui nous est présenté est-elle intégré n'est-elle pas intégré. Je voudrais également rappeler que puisque vous visez un taux d'emploi d'amélioration du taux d'emploi des seniors une amélioration de 10 points du taux d'emploi des seniors d'ici 2032 rapporterait 2% du PIB et 50 milliards de richesse selon des économistes. Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur enfin une augmentation raisonnable de la masse salariale des fonctionnaires rapporterait 3 3 milliards. Quant à l'hypothèse d'un taux de chômage à 4 et demi pour 100, à partir de 2027, cette hypothèse se traduirait par un excédent de 20 milliards de l'Unédic.

Il va falloir commencer à émettre du vôtre, messieurs les Ministres cela démarre mal avec Sertic cet article liminaire qui est censé nous présenter les prévisions budgétaires sur lesquels vous fondez l'ensemble de cette réforme et il est déjà en soi un manque de respect pour notre assemblée, que vous nous proposez est contestable. Nous aurons l'occasion d'en discuter mais ce qui est problématique, c'est que vous l'par des prévisions contenues dans un texte qui a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale qui n'a donc jamais été validée par le Parlement. En d'autres termes vous affichez une colonne de chiffres issus d'un texte qui n'existe pas et vous attendez que nous le prenions pour argent comptant. Cela en dit long sur la considération que vous portez et que vous avez pour le Parlement, et pour le Sénat en particulier à l'Assemblée à l'Assemblée nationale vous avez osé répondre à notre collègue Jérôme Guedj, que vous n'aviez pas pas à rendre de comptes ni sur les canaux, ni sur la manière dont vous faites les prévisions. J'espère que vous êtes venus devant nous dans dans d'autres dispositions d'esprit car nous n'aurons de cesse et comptez sur nous, aujourd'hui et jusqu'au 12 mars, de vous demander des comptes c'est une c'est notre prérogative de parlementaires de contrôler le gouvernement, ne vous en déplaise. C'est aussi notre devoir de la clarté dans de maîtres de la clarté dans un débat qui a souffert de beaucoup d'enfumage et qui intéressent pourtant l'ensemble de nos concitoyens depuis des mois vous crier sur tous les toits que l'enjeu est de sauver notre système de retraite par répartition et que les Français devront tous sacrifié 2 années de leur vie pour cela. Alors la moindre des choses c'est de nous dire ce que nous allons vraiment payer en faisant ces sacrifices parce que vos estimations sans même parler de ce fameux projet de loi de programmation fantômes semble très artificiel le déficit que vous annoncez et très largement gonflée. Ils se basent notamment sur une poursuite de l'allongement de l'espérance de vie qui stagne. Pourtant, 2000 depuis depuis 2014 ou des prévisions de recettes partir du Mans faible par exemple sur les salaires des fonctionnaires. En conclusion, je vous dirai simplement ceci, et il y a un langage de vérité, arrêter les faux-semblants il ne venait pas nous parler de réforme de progrès social ou de justice tous 2 également absent de ce texte. Donnez-nous les comptes tous les comptes et rien que les comptes mais les vrais et peut-être que dans ces conditions, le débat se passera mieux qu'à l'Assemblée. Monsieur le président. Messieurs. Les ministres. Chers collègues je dans la même veine que mes 2 précédents. Collègues. Voilà un texte qui est présenté de manière fort. Curieuse, d'autres ont dit cynique voire machiavélique. Loi de financement donc anti-car recevabilité. On n'avait pas d'étude d'impact. Donc vous avez des fiches d'évaluation. Voté en commission mais ce qui a adopté en commission le figure pas dans le texte en séance publique. l'assemblée ne votent pas le texte. Hé ben on retrouve l'entièreté du texte telle qu'il a été conçu par le gouvernement, c'est quand même une curieuse procédure. Même si on veut être hyper responsable et sage comme on est ici dans cette assemblée. Il faut quand même être conscient qu'nous piétinent et qu'on nous abîme alors si c'est ça le mi-Carême risque ce n'est pas vraiment ma conception et c'est pas celle si j'ose dire de ce camp-là ici. Dans l'hémicycle. C'est un peu curieux qu'on fasse ici, matin et soir l'éloge des deux chambres. De l'indépendance et que, au nom d'une certaine sagesse et de l'art de gouverner. Eh bien nous acceptions. Ceux cela ce texte, c'est l'architecture même l'architecture financière de votre projet l'accepter. Ou le rejeter le rejeter, c'est faire tomber tous les autres textes tout le texte. Et là c'est vrai c'est. Le PIB se gagner ici ou là quelques centaines de millions, ce n'est pas bougé au motif que nous devons préserver l'attractivité et la compétitivité du pays et qu'il ne faut donc pas augmenter les impôts

projet portant sur. Le système et l'architecture faut conclure qu'est ce qu'il fallait penser, c'est uniquement de nouvelles recettes que vous refusez d'envisager. C'est un classique du genre à chaque réforme des retraites on dramatise la situation pour expliquer qu'il faut remettre en cause tous les acquis sociaux de ce pays. Et là le cette affaire, c'est de la même veine. Vous annoncer à leur manque de chance, le corps a quand même énormément relativiser en disant que les le système était maîtrisé que certes il pouvait y avoir un déficit mais que ce déficit était quand même si je puis dire aisément, n'exagérons pas mais facilement qu'on blâme. Mais surtout quand on regarde de près vos hypothèses. Une des clés. De l'accroissement du déficit. C'est la baisse de la participation de l'État. Et ça vous ne le dites pas aux français. Vous ne dites pas aux français. Que vous n'allez cause créé aucun poste de fonctionnaire, jusqu'en 2027. Certes les 15.000 postes du Ségur sont prévues dedans mais rien d'autre. Pas de poste de prof. Pas de poste de d'infirmières supplémentaires. Pas d'amélioration du système de justice. Deuxièmement ce n'est pas une petite perte. Les syndicats estiment que dès la fin du quinquennat. C'est 3 milliards d'euros en moins et on tombe à 4 milliards de déficit et à l'échéance 2037 2040 c'est entre 9 et 18 milliards du simple au double. Cette question est centrale. Premièrement l'état, le pays a besoin de fonctionnaires et deuxièmement qu'est-ce que vous allez faire geler le point d'dit c'est d'ailleurs écrit dans les les estimations du corps gelé le point d'indice, ce qui veut dire que les fonctionnaires perdront d'ici 2035 29 37 8 % de leur pouvoir d'achat. Ah évidemment inflation comparables pendant que ceux du privé verront leur pouvoir d'achat théorique augmenter de 12. La Moindre des choses. C'était le parallélisme des trajectoires ou sacrifier l'avenir de la fonction publique sans dire aux Français. Et vous, vous vous utilisez ce critère pour gonfler hein. Merci monsieur le président. Nous allons discuter d'un article liminaire, alors qui dit article liminaire dit loi de finances. C'est bien là que le bât blesse. Nous avons bien entendu hier Madame la rapporteure générale nous expliquer que. Le fait qu'on puisse parler de retraite dans le cadre d'une loi de finances de la dérangeait pas. C'est vrai que d'un point de vue extrêmement technique, dans la mesure où nous allons reporter vous comptez reporter l'âge de la retraite. Ça va faire. Des dépenses. En moins et donc ça va améliorer les comptes publics. C'est bien là que le bât blesse aussi. Vous avez pris, messieurs les ministres, le gouvernement a pris des engagements. Pour abaisser le niveau de la dépense publique. La part des retraites dans les dans les dépenses publiques et particulière, il est important hein. Et donc il vous a semblé que finalement le plus simple c'était d'aller taper dans les retraites mais taper dans les retraites, ça veut dire quoi. Ça veut dire s'il est question de faire rentrer de l'argent immédiatement dans les caisses de l'État. Ça veut dire forcément. Pénaliser des gens qui sont prêts à partir à la retraite entre 6 mois et 2 ans. Et ces gens-là ils ont déjà plus de 40 annuités de cotisation il travaille depuis 41 42 ans et donc c'est finalement à eux que vous allez expliquer. Qu'ils doivent être améliorés par leur sacrifice le sacrifice de leur travail, qu'ils doivent améliorer les comptes publics. Tout ça c'est des débats bien compliqué. Et vous pourriez penser que finalement les tombes pas n'étant pas rompu à tous ces débats. Ces salariés ne comprennent pas. Messi, Messi, Messi, ils ont parfaitement compris. C'est bien pour ça qu'ils sont extrêmement défavorables et qu'ils seront dans la rue mardi prochain. Monsieur Assouline. Nous sommes donc à l'Arctique liminaire. Et dans ce débat. Nous sommes aux préliminaires. On va dire que. Ça commence bien. Tout le monde voulait un débat. Apaisé où chacun peut expliquer les choses, faire des démonstrations. Les autres, écoutez. Nous enrichir tous parce que on apprend des interventions des uns et des autres et de ce fait, on est claire aussi l'opinion. Et donc. Je pense que ce débat commence très bien. Et si cette année un article liminaire, il nous dit tout. De l'état d'esprit de cette réforme. Vous pensez bien que la question des retraites. Taraude tous les politiques et tous les citoyens, les jeunes en particulier depuis plusieurs années. Parce qu'il voit bien. Que il y a pas que la démographie qui a bougé. Mais le monde du travail lui-même. Est bouleversé. Toutes les relations du travail et personne ne sait d'ailleurs dans 10 ans. Quelles seront ses nouvelles relations et l'état. De de de la production de la façon de produire. Et donc, y compris des mécanismes sociaux nouveaux qu'il faudra inventer avec ces révolutions technologiques et puis il y a aussi le réchauffement climatique qui bouge quasiment tous les paramètres que nous connaissions il y a encore quelques années et là aussi les projections et les impacts sur le travail sur. La pénibilité sur tout un tas de domaines qui touchent en conséquence en retraite ne sont pas évalués et le Parlement devrait servir à ça et on vient ici nous dire que à 30 ans, ça va être déficitaire. Sans élément de discussion plus globale qu'une réforme financière et c'est pour se on dans cet article liminaire, tout est dit. C'est une vraie conclure comptable et pas une réforme sociale. Monsieur le. Le président, chers collègues, je pense que c'est important que nous le soulignons au début de, de, de notre débat nos échanges. il y a un vrai souci de de méthode depuis le début avec ce gouvernement. Je pense qu'il vous honorez-vous aussi à droite de le signaler. Je pense que on parle quand même d'un sujet d'une réforme qui touche au coeur de notre pacte social qui peut pas être discutée dans un délai aussi contraint aussi restreint avec une volonté brutale de la part du gouvernement de piétiner nos droits en tant que parlementaire de pouvoir légiférer, de pouvoir discuter d'avoir le temps de discuter, d'échanger sur des choses qui engage plusieurs générations. Ça en dit long quelque part sur votre politique. Monsieur le ministre, et à travers ce gouvernement. Sur sur la violence finalement de cette réforme, à travers vous violenter les Français à travers cette réforme vous violenter le Parlement et ainsi la démocratie parlementaire avec avec cette, cette procédure, avec d'ailleurs avec la complicité de la droite sénatoriale puisque depuis le début le dépôt de nos amendements. J'ai regardé. Nous en sommes à 1000 amendements rejetés sur des motifs alors que auparavant la plupart d'entre eux été acceptée dans les les précédents Plfss a été ça dit par par des collègues à juste titre- parce que moi-même j'en avais déposé dans les précédents était accepté. Ils ne le sont pas cette fois-ci ça monte quand même que, main dans la main. Vous avez également cette volonté de nous empêcher de débattre réellement d'ailleurs sur le fond accepter nos amendements et nous le ferons parce que le prétexte qu'il est employé, c'est de dire que ça ne porte pas sur l'application d'une loi de financement de la Sécurité sociale mais madame la présidente de Roche. C'est l'ensemble du PLFR. Qu'il faut déclarer recevable parce que c'est l'ensemble de ce projet qui ne correspond pas justement à une loi de financement de sécurité sociale. C'est pour ça que le le gouvernement vous feriez mieux de d'avoir un petit peu le courage de faire une loi ordinaire

Cet article minime Miller votre bien votre impératif d'équilibre des comptes publics, mais pour notre part, aborder une réforme des retraites. Uniquement sous un aspect financier. Ce n'est pas une bonne chose, s'est montré un très mauvais message à nos concitoyens. de retraite, c'est le résultat d'une vie de travail pour une grande majorité de nos compatriotes, c'est eux qui ont passé toute leur vie au travail et qu'est-ce qu'ils recherchent une meilleure qualité de vie pour leur retraite. Vous justifiez votre réforme sous le. Le le déficit par la démographie. Je voudrais quand même rappeler quelque chose, ce n'est pas que la démographie certes elle est là mais c'est aussi toutes les exonérations des charges sociales, c'est aussi toute la réduction du nombre de fonctionnaires ainsi que leur niveau de rémunération qui assèche les les les financements des retraites, ça aussi ça doit être pris en compte. Ensuite, le comité d'organisation des retraites a bien dit 2% du PIB et le retour à l'équilibre en 2050. Je crois qu'effectivement ce déficit, il est tout à fait supportable 2% du PIB. Surtout quand on pense que le le la retraite comment c'est important pour dans camp de citoyens 2% de PIB. Qu'est-ce que c'est en mais bien d'autres argent à d'autres moments. Je crois qu'il est important que l'État prenne ses responsabilités et puis moi j'aimerais avoir une autre information. Parce que on ne mesure absolument pas mais vous le faites toujours avec vos lois. L'aime pas que ça peut avoir sur d'autres sujets, induits de certains dispositifs de cette report forme sur les finances publiques sur le chômage, sur le RSA sur la c'est santé publique je voudrais vraiment que nous puissions vraiment évaluer financièrement cela aussi. Dernière orateur inscrit madame de La Gontrie et ensuite je donnerai la parole monsieur le ministre Attal. Merci, monsieur le Président, sur cet article liminaire, il faut quand même être conscient qu'il vise donc à entériner une réforme paramétrique des retraites qui répondrait selon vous un impératif d'équilibre des comptes publics. Ils présentent des agrégats qui doivent être comparés selon vous à ceux d'une loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 mais il n'y a pas de loi de finances publiques qui a été votée par le Parlement, puisque vous le savez le gouvernement a préféré ne pas faire voter ce texte par l'Assemblée, par peur de le voir rejeté. le gouvernement aujourd'hui et sans règles ni boussole concernant sa stratégie de finances publiques mais avec des déficits publics, il a creusé avec des cadeaux fiscaux aux entreprises et aux plus aisés. Nous le savons très bien, donc vous n'avez pas de vision de long terme. Vous vous ménager un chemin budgétaire à coups de dans notre protection sociale et vous prétendez aujourd'hui utiliser la réforme des retraites pour combler ses déficits vous donner ainsi des gages à l'Union européenne évidemment, mais on le voit bien aujourd'hui ce souci des finances publiques ne se situe pas en réalité vous devriez en être conscient. Au niveau du système des retraites. Il est en réalité ce système de retraite. Il souffre d'un problème de recettes mais sur lequel vous refusez de vous pencher et c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article qui ne se réfère aucune loi de programmation des finances publiques. Contrairement à sa rédaction et qui ne sert qu'à sous-tendre une stratégie de sauve qui peut désordonnée du gouvernement qui prétend ainsi sacrifier une partie de notre système de retraite dans la poursuite d'un objectif qui ne le concerne pas. Monsieur le Président rapidement puisqu'on va poursuivent la discussion à l'occasion des. Amendements de suppression de cet article liminaire mais pour répondre à quelques points. D'abord sur la question du déficit. J'ai entendu l'intervention de monsieur. Savoldelli. Mais qui à la fin si on vous suit revient à dire qu'on déplace en déficit. On déplace le déficit du système de retraite vers d'autres branches de la Sécurité sociale, ce qui évidemment pas notre objectif, notre objectif c'est de réduire les déficits, pardon les déplacements d'une branche à l'autre mais en les réduisant en prenant des mesures et en réformant notre système. Le fait est qu'il y avait 12 millions de pensions à payer chaque mois en 2002 et qu'il y en aura 30 millions à payer en 2030 ça a doublé sur une génération parce qu'on vit plus lentement, plus longtemps et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais entre temps vous n'avez pas non plus un doublement du nombre d'actifs, même s'il a augmenté. Et donc vous devez forcément prendre une mesure pour équilibrer le système, sinon vous ne pouvez plus payer les pensions de retraite. Et donc à partir de là il y a une proposition et je comprends que c'est la ligne de la gauche qui est d'augmenter les impôts. Ça a le mérite de la clarté, c'est votre proposition, augmenter les impôts. On avait beaucoup d'discussion là-dessus à l'Assemblée nationale. Ah non non non on viendra dans les discussions sur les amendements mais à l'Assemblée, c'était pas les riches ou alors on considère que un retraité à 1500 euros et riche. Parce qu'en l'occurrence à l'Assemblée. Je parle de l'Assemblée nationale. Je parle du débat que nous avons. Mais oui, et c'est pour ça que je dis qu'on aura la discussion sur vos amendements mais On aura la discussion sur vos amendements qu'on verra et vous verrez que parfois. Derrière un amendement qui prétend taxer des très riches. Bah en fait. Le diable est dans les détails et souvent ce sont des Français de classe moyenne qui sont touchés par les amendements qui prétendent taxer les riches. 2ème, chose que je voulais dire sur les déficits. J'ai eu le sentiment dans certaines interventions que un déficit à 13 milliards cinq ça serait rien enfin c'est pas une paille, 13 milliards Est pas une paille. C'est-à-dire c'est 2 fois le budget du ministère de la justice. C'est l'équivalent de ce qu'on dépense pour les APL. C'est quand même majeur et si j'ai entendu, j'ai entendu certaines interventions dire. 13 milliards cinq finalement ça pourrait être beaucoup plus. Effectivement, ça peut toujours être beaucoup plus mais du coup, vous me permettrez, vous me permettrez de de tirer le fil de ce discours que vous avez tenu. Jusqu'à la fin ça veut dire que vous reconnaissez que vous validez que vous soutenez la stratégie économique de ce gouvernement et de notre majorité, parce que si on n'a pas un déficit plus important. C'est pourquoi c'est pas ce qu'on a créé 1.500.000 emplois depuis 5 ans et 1.500.000 emplois depuis 5 ans, c'est 25 milliards de cotisations sociales en plus pour notre système de retraite. Donc par ce discours vous valider nos mesures. La création de la flat tax, la suppression de l'ISF les allégements de cotisations, la baisse de l'impôt sur les sociétés des entreprises, c'est ce qui a permis à l'activité économique de se développer, c'est ce qui nous a permis d'avoir une augmentation des créations d'emplois d'un million cinq et donc des recettes en plus pour notre modèle social. La dernière chose. La dernière chose à laquelle je veux répondent, c'est madame Monge. Vous êtes intervenu sur la question des mesures sociales. Et je vous remercie de l'avoir fait. D'abord, vous avez dit finalement, le fait de maintenir un âge de départ à 62 ans pour invalidité n'est pas une mesure sociale puisque c'est le la situation actuelle. Sauf que la situation actuelle dans le code de la sécurité sociale, il est dit que l'âge de départ pour invalidité est le même que l'âge légal de départ. Et à chaque fois que l'âge légal de départ a été reculé, y compris en 2010 lors de la réforme Woerth. L'âge de départ pour invalidité a été reculé aussi. Donc ce que nous faisons dans ce texte, c'est que nous créons un âge de départ anticipé pour les départs en invalidité et effectivement il y a un coût de 3 milliards d'euros. Mais je vous remercie d'avoir mis en avant la question des mesures sociales de cette réforme. Parce que j'ai été regardé. J'ai été regardé la le budget des mesures sociales des précédentes réformes des retraites. Réforme des retraites d'Éric Woerth en 2010 mesures sociales autour d'un milliard 5. Réforme des retraites de Marisol Touraine, en 2014 très bonne réforme. Coût des mesures sociales 4 milliards. Réforme des retraites de ce gouvernement en 2023 mesures sociales 6 milliards d'euros. Ça veut dire que les mesures sociales contenues dans cette réforme sont plus importantes en montant que celles qui étaient contenu dans les deux précédentes. Réforme des retraites confondus. Ça dit l'ampleur des mesures d'accompagnement que nous prenons précisément pour répartir l'effort de la manière la plus juste possible dans le cadre de ce texte. Mais nous aurons l'occasion d'en parler dans le pendant les les jours à venir.

Cette réforme des retraites est porté dans le cas d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, comme nous l'avons souligné hier avec madame la rapporteure générale pour une seule raison, c'est que l'ensemble des mesures que nous proposons, ont un impact sur les comptes sociaux et que ça. Justifié et légitime. Ce dispositif et le choix de ce véhicule législatif. Pour ce qui concerne l'avis du Conseil d'État. J'ai dit tout à l'heure et je le répète. Pour être sûr d'être entendu que. Il n'y a pas d'avis rendu par le Conseil d'État sur un projet de loi de finances ou un projet de lorsqu'on la sécurité sociale, qu'il y a une note de synthèse et j'ai rappelé dans quelles conditions. J'ai rappelé monsieur le sénateur Assouline dans quelles conditions cette note de synthèse et consultable par un certain nombre de de parlementaires otite de leur fonction de contrôle. C'est la règle, elle peut être respectées et si parmi vous il y en a qui sont investis de ses fonctions. Ils sont litres de se rapprocher du secrétariat général du gouvernement pour la consulter dans les mêmes conditions que cela a été fait précédemment. Pour en venir à l'interpellation. Plus que la question de monsieur le sénateur fera ça. Je voudrais simplement vous dire, Monsieur le Sénateur que. Sur les 3 points que vous avez évoqué, vous avez parfaitement raison. La difficulté d'absence de conventions de coopération fiscale, sociale et en particulier social entre la France et certains pays de résidence de Français installés à l'étranger. La difficulté du de devoir choisir un pays pour lequel il y a une forme de de récupération de transfert des droits et enfin la disposition de la difficulté liée au au salaire de référence. Aucune des dispositions qui pourraient répondre à ces 3 problèmes ne peut trouver sa place dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui soit rectificatif ou non puisque toute relèvent de conventions de coopération entre la France et les États concernés. C'est un chantier assez titanesque puisqu'il y a autant de chantiers à ouvrir que de pays de résidence. Mais j'ai eu l'occasion de le dire un certain nombre de parlementaires. Élus des Français de l'étranger, député ou sénateur, je pense que c'est un chantier que nous devons ouvrir. Je pense même que plus nous l'ouvrirons de manière collective partagée entre les des chambres et les différentes forces politiques du pays et mieux ce sera. Avec à chaque fois un horizon qui ne peut pas être très proche puisque cela juste cela nécessite la discussion de conventions internationales et ensuite l'adoption de 2 projets de loi permet ou de propositions permettant la ratification des dite de convention mais rendez-vous est pris pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Merci nous allons passer maintenant à l'examen de 62 amendements en discussion commune. Ils sont tous identiques. Ils portent tous sur la suppression je donne la parole à Madame, la présidente, Éliane Assassi. Pour le premier amendement. Merci. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues. Donc l'article liminaire de ce texte. Prévoit un solde public de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. En déficit de moins 0 8 % soit le même chiffre que celui adopté dans dans la loi de financement de la Sécurité sociale. En décembre dernier, ce qui n'est pas vieux hein si c'est. Selon l'exposé des motifs de l'Arctique je cite la prévision retenue est quasi identique à la prévision sous-jacente à la loi de finances pour 2023. En effet, elle n'en diffère qu'au titre de la réforme des retraites dont l'impact pour 2023 est faible et proche du montant provisionné lors du projet de loi de finances, fin de citation. Dès lors cet tactiques renforce notre argumentation qui vise à critiquer l'utilisation d'une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, puisque les effets pour 2023 son je récite quasiment identique en effet l'impact de la réforme des retraites sur les finances publiques en 2023 est estimé à seulement 400 millions d'euros sur un budget total de la sécurité sociale de 722 milliards d'euros, soit une évolution de l'ordre de 0, 0 5 %, c'est-à-dire rien du tout. À titre de comparaison, la loi de financement pour 2023 à rectifier les comptes de 2022 pour un écart de 19 milliards d'euros par rapport donc aux prévisions. On peut donc largement penser que les écarts entre les prévisions voté pour 2023 et les résultats réalisés seront largement plus important que ce qui justifie cette loi de financement rectificative, je le répète 400 millions d'euros. En réalité. La vérité est ailleurs, comme dirait l'autre. Le gouvernement a fait le choix de ce véhicule législatif uniquement. Dans un but pour lequel il n'est pas fait. J'y vois même de l'opportunisme politique pour conserver un usage futur d'un recours à l'article 49.3. De la Constitution et imposer des délais de dépôt de débats suffisamment resserré. Pour éviter une mobilisation sociale copains dur et qui sera manifestement très grande le 7 mars prochain. Un amendement 126 madame pour ces mon. Merci monsieur le président. Mais quand même, préalablement je tiens à dire à monsieur Attal, que je suis très inquiète pour notre maîtrise des comptes publics et le fait qu'il vous soit confiée. Vous appelez, mesures sociales, le maintien des droits mais sur le plan financier, ce maintien n'est pas un coût supplémentaire. Je le maintiens moi il ne participe pas aux gains de la réforme, certes, mais il n'est pas un coup ce n'est pas une mesure donc vos mesures, c'est 3 milliards, c'est-à-dire 3 milliards par rapport à 18 milliards. C'est, voilà la réalité. Bien alors au cours du 1er mandat d'Emmanuel Mâcon les nouvelles baisses d'impôts essentiellement au profit des grandes entreprises et des contribuables les plus fortunés. d'ISF la flat tax ont amputé le budget général de l'état de 50 milliards d'euros de plus par an. Selon Bercy, même le choix de procéder à une nouvelle suppression de recettes des comptes publics que représente la cotisation sur la valeur ajoutée CVAE. Dont les recettes annuelles s'élèvent à plus de 12 milliards d'euros et qui sont liés aux quand même aux chiffres d'affaires des des grands groupes, ils laissent le choix du gouvernement de creuser le déficit et justifiera l'austérité des dépenses publiques auprès de la Commission européenne. Il en va de même pour le faible, déficit du système de retraites sur le budget de la Sécurité sociale. Cela ne réside Topor d'un défi déséquilibre démographique non anticipée mais du démantèlement depuis 2010 du fonds de réserve pour les retraites du tarissement délibérée des ressources et des politiques austéritaires. À commencer par la fonction publique au nom du nombre des fonctionnaires et du gel du point d'indice. Programmé. C'est pourquoi par cet amendement. Nous proposons la suppression de cet article liminaire. ville de votre vision étriquée des objectifs financiers de votre coup gouvernement au profit de cette contre-réforme des retraites. Monsieur le président Gontard présent de l'amendement 127. Merci monsieur le président. Par cet amendement de suppression. C'est tout l'équilibre budgétaire que nous réfutons

gel du point d'indice de la fonction publique et plus largement une politique malthusienne en termes d'emplois publics imputation de la dette Covid aux comptes sociaux plutôt qu'au budget de l'État. Ce déficit des caisses de retraite, c'est avant tout votre bilan et évidemment vos choix budgétaires, mais c'est également de votre coalition de droite avec la réforme Fillon, le gouvernement Jospin avait été prévoyants en instituant en 99 le fonds de réserve pour les retraites qui aurait dû être dotée en 2020 de 65 milliards d'euros pour faire face justement à la diminution du ratio actifs travailleurs sans pénaliser les travailleurs. Rappelons que ce ratio est temporaire que nous sommes dans une période de bosse démographique due à l'arrivée massive à la retraite de la génération du baby-boom. Ces réserves du FFR devait permettent de combler les déficits des caisses de retraite pour toute la décennie 2022 1030 mais les multiples sources de financement du FFR ont été rabotées par la réforme des retraites de 2010 de messieurs Woerth et Fillon aujourd'hui nous payons cette incurie. Nous payons votre dogmatisme anti-impôt. Nous payons la vision économique éculée des droites. Pas étonnant de vous retrouver les majorités présidentielles et sénatoriales main dans la main dans ce dossier, vous êtes coresponsable de la situation actuelle et pour réparer vous réserves heures c'est toutes les Françaises tous les Français que vous voulez faire payer avec cet impôt sur la vie de deux ans. supprimant donc cet article, nous vous proposerons tout au long de la première partie de ce débat des solutions de recettes alternatives pour rééquilibrer nos caisses de retraite et nous vous montrerons par A plus B que bien d'autres solutions sont sur la table et au moins la décence pour la suite de nos débats

Merci monsieur le président. D'abord je voudrais remercier la présidente de Roche de ces explications détaillées sur les. Recevabilité qui souligne à quel point le gouvernement fait preuve d'une ruse de procédure en imposant ce débat dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale qui ne permettra pas l'entièreté du débat sur des sujets essentiels, je pense notamment à la question de l'index senior entre autres ma 2ème remarque c'est pour dire à Monsieur le Ministre que je n'ai pas sa compétence et sa connaissance et qui hier j'avais confondu avis avec note de synthèse s'agissant du Conseil d'État. Mais Monsieur le Ministre sans compétence et sans connaissance. J'ai une très bonne connaissance des Français et je peux vous dire que le secret en matière financière sème toujours le doute et fait le lit de la démocratie. Je vous demande donc à nouveau de publier pour tout le monde. La note de synthèse de la rende. Plutôt que de la laisser uniquement à l'intention des parlementaires qui ont accès. Ma dernière remarque sur cet article liminaire. Pour 400 millions d'euros de mouvements, nous allons prendre 2 ans de la vie. de nos concitoyens pour 400 millions. Nous ne pouvions pas attendre soit un projet de loi de finances classique, soit un texte ordinaire comme ça aurait été nécessaire. Il convient de supprimer, d'autant que d'autres hypothèses sont possibles. Imaginez une nouvelle crise Covid imaginer des canicules qui vont venir modifier tout ça figure dans une réforme paramétrique puisque vous faites le choix d'une réforme paramétrique. Je veux vous dire que 2 ans de la vie des gens, ça n'est pas un paramètre, c'est une question fondamentale.

Il dit d'abord que par l'évolution très marginal. Des des chiffres budgétaires. Le véhicule législatif ça a été dit et largement un prétexte pour limiter le temps de débat. Il dit aussi qu'il n'y a aucune ressource financière nouvelle. Et Monsieur le Ministre, même si vous pointez tel ou tel amendements de l'Assemblée nationale, la réalité c'est qu'il n'y a aucune ressource nouvelle sur les revenus du capital sur les plus riches sur les grandes entreprises, et notamment sur les superprofits. Il ne dit pas non plus. Il lui manque une ligne, il y a bien un impôt nouveau dès cette année 2023 un impôt de 3 mois. De vie sur nos compatriotes qui sont nés dans le dernier tiers de l'année 1961, cette réforme elle est particulièrement brutal tous les travailleurs qui sont nés dans les années 60 et cela commence par ceux qui sont nés à partir du 1er septembre 1961 cette ligne elle doit aussi être ajoutés à votre tableau et puis ensuite il y a un problème de légitimité. Cette réforme elle est comptable et elle s'inscrit dans une trajectoire des finances publiques qui n'a aucune légitimité démocratique puisqu'elle n'a pas été votée par le Parlement. Il y avait une phrase sibylline dans le projet de loi de programmation des finances publiques qui était la soutenabilité de notre trajectoire reposera sur les réformes structurelles engagées en réalité les réformes structurelles engagées, c'est celle que vous nous présentez aujourd'hui cela ne s'appuie pas sur le vote du Parlement. Cela. Vous mettez donc la charrue avant les boeufs, faites d'abord adopter une loi de programmation des finances publiques et ensuite nous parlerons de loi financières pour les années qui viennent. Merci. L'amendement 341 présenté par Madame. Merci monsieur le président. Hein, mes chers collègues. Si j'ai bien entendu hein. Monsieur le Ministre tout à l'heure vous avez a. Dit que le le déficit était bien moindre que prévu grâce. Au au fruit de votre politique. Du coup, une demande pourquoi, mais pourquoi cette réforme. Il suffisait donc d'attendre un peu, tout simplement. Et pourtant, cet article. Entérine financièrement une réforme injustifiée qui relève des seuls choix du gouvernement. Ceci afin d'afficher une réduction globale du déficit qu'il a lui-même aggravée par les cadeaux fiscaux généreusement distribué ces dernières années. d'autres solutions existent. Qui imposent. Il est vrai, de se poser la question des recettes du système. Il convient donc de supprimer cet article. Qui ne traduit nullement une nécessité mais bien une vision idéologique, celle de faire des réformes toujours au détriment de toute justice sociale. Merci monsieur le président. Oui sur cet amendement, donc qui vise à supprimer cet article, je ne vais pas revenir sur les arguments que mes collègues ont emporté de ce côté-ci de l'hémicycle et qui auquel je je je je m'associe totalement mais je voulais revenir particulièrement sur l'ajout de 750 millions d'euros pour le rehaussement de l'Ondam pour sauver ossements de l'Ondam qui serait en particulier. Consacrée à l'hôpital public mais il n'est nettement insuffisant nettement insuffisant si on tient compte. De l'inflation, ils baissent que même par rapport à 2022, de 5,2% alors insuffisant. nos hôpitaux que vivent pardon nos hôpitaux publics ici comme ailleurs dans le Calvados, mon département comme ailleurs sur le terrain, nous en voyons les effets très concrètement c'est-à-dire que que ce soit au CHU de Caen à l'hôpital de fadaises à l'hôpital de Lisieux à l'hôpital. de proximité. Les hôpitaux de proximité, pardon, les besoins en personnel sont alarmants. Beaucoup de ces établissements ont été contraints de fermer provisoirement heureusement le service des urgences. D'autres ont été contraints de fermer d'autres services, et cela n'est pas acceptable ni pour nous les parlementaires mais surtout pour nos concitoyens. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise. À supprimer l'article liminaire car il entérine financièrement une réforme paramétrique des retraites injustifiées et injuste. Celle-ci répond à un impératif d'équilibre des comptes publics. À la suite d'une politique intensive de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Fin de la CVAE. Et aux ménages les plus riches. Suppression de l'ISF, création de la flat Mais aussi d'un transfert de la dette. 19. Ce décompte de la protection sociale. Or, d'autres solutions existent, elles exigent de me poser la question des recettes du système question absolument taboue par le gouvernement. Pourtant les les exonérations de cotisations sociales dont certaines sont sans aucun effet notable sur notre économie coûteront à la branche vieillesse 18,9 milliards en en 2023, soit un peu plus que les 17 7 milliards d'euros que le gouvernement cherche d'ici 2030 à travers sa réforme. D'autant que cette 17. 7 milliards escomptés ne tiennent pas compte des coûts induits du report à 64 ans de l'âge légal du départ à la retraite pour l'assurance chômage et les minima sociaux.

Tout d'abord l'indigence de l'annexe explique il tête explicatives jointes à ce projet de loi peut nous laisser sans voix puisque. Le législateur est sciemment mal informés. Pourquoi. Qu'avez-vous à cacher. Publié justement cette note de synthèse comme ça a été bien rappelé par mes collègues. Pourquoi avez-vous peur de de la transparence. Nous attendons donc toujours plus de précisions. Pourquoi. Prévoyez-vous une diminution de 1 11 % de la masse salariale des fonctionnaires. Est-ce à dire que ceux-ci connaîtront une paupérisation relative et absolue sans précédent. Le corps souligne dans son rapport les effets d'un gel du point d'indice jusqu'en 2027 et de l'augmentation très réduite qu'il connaîtrait à partir de cette date. Pourquoi. Présentez-vous certains déficits en euros constants et le PIB en euros courants. Ce qui empêche toute comparaison juste. Autre question importante pourquoi. La part des rémunérations des agents des collectivités territoriales diminue dans l'ensemble des rémunérations alors que leur taux de cotisation est supérieur à celui d'autres régimes. Pourquoi n'avoir pas pris en compte une augmentation du taux d'emploi des seniors sur laquelle vous fonder quelques espérances, pourquoi les femmes ont-elles dans vos prévisions. Un taux d'emploi inférieur de 8% à celui des hommes, alors que l'égalité salariale est censée être l'une des grandes causes nationales. Au final, le déficit que vous mettez en avant pour justifier cette réforme ne viendrait-il pas des hypothèses factice outre. Que vous avez fourni au corps d'où nous saluons par ailleurs le travail dans ces conditions. d'ailleurs, c'est toujours la même méthode avec vous vous diminuer. Les cotisations sociales, donc le chien à la rage et comment on règle c'est pas on les on les rois augmentant non c'est un allongement sans cesse la durée de départ de la âge légal. Puis, merci Bernard de La Gontrie, Merci monsieur le président. Selon les prévisions de la Commission européenne publiées récemment sur les 20 pays de la zone euro, la France est celui où l'investissement reculera le plus en 2023. C'est pour cela qu'au lieu d'engager cette réforme injuste et inutile. Vous feriez mieux de vous occuper de l'état de la France de son industrie et des investissements. Vous dites vouloir faire grâce à la réforme, une économie de 18 milliards dont les 2 tiers. S'il y a qu'un seul ministre et qu'en plus à nos collègues lui parle. Ça va être compliqué, enfin sauf s'il. dans les 2 tiers seront payés par les femmes. Mais combien d'argent avez-vous gaspillé en ayant pas renégocier le prix de l'électricité sur l'année 2023 ce sera l'lors de 30 à 50 milliards. Vous approuve ouvrirez ainsi les l'industrie française. Les commerçants, les TPE, les PME. Car telle est bien le sujet. Cette année, réduire le prix de l'énergie afin que les artisans, les TPE, les PME continuent à investir et enfin parlons du rapport du COR, qui a été peu évoqué jusqu'à présent, vous le savez, les résultats du rapport ne valide pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraites et il précise, à plus long terme malgré le vieillissement progressif de la population française. La part des dépenses de retraites dans la richesse nationale serait stable ou en diminution. Voilà. Monsieur le Ministre pourquoi nous considérons que cet article liminaire qui par ailleurs n'est appuyé sur aucune loi de programmation des finances publiques mais je l'ai évoqué tout à l'heure doit être supprimé. Monsieur Redon Sarah il. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement cet article liminaire nous souhaitons. Qu'ils soient supprimées parce qu'il entérine financièrement une réforme que nous visons injustifiée et injuste. Elle est injuste avant tout. Car comme vous le faites depuis déjà plus de 5 ans, Monsieur le Ministre. Vous n'avez de cesse de faire supporter les efforts non pas aux plus riches. Mais à ceux de nos concitoyens les plus modestes. Pour votre gouvernement. Les plus riches doit être épargné de tout effort qui soit fiscal ou de toute solidarité. Fin de l'ISF, fin de la CVAE flat tax sans doute encore d'autres cadeaux que vous avez en réserve pour demain. Hors de question pour vous de vous interroger sur des recettes nouvelles ou plutôt, même sur des recettes qui pourrait redevenir des recettes, je veux parler. D'exonérations qui, bien que très coûteuse. Pour les comptes. La branche vieillesse ont des efforts en matière d'économie qui reste à démontrer. Et nous aurons tout au long de ces débats à l'occasion de vous démontrer que les économique vous escomptez avec votre report à 64 ans. Risquent de se reporter très défavorablement vers l'assurance chômage vers les vers les minima sociaux. Merci Merci Monsieur le Président. Cet amendement donc de suppression. De l'article liminaire, qu'un. Mais vous est proposé car il entérine financièrement une réforme paramétrique des retraites qui préempte 2 ans de la vie des Français. Une réforme donc injustifiées et injuste. Les 17 7 milliards escomptés ne tiennent pas compte des coûts induits du report à 64 ans de l'âge légal. La réforme en augmentant l'âge de départ dès 2003 provoque des dépenses supplémentaires par l'assurance chômage, les aides sociales ou encore l'assurance maladie de salariés sur 5 ne sont déjà plus en emploi lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite, ils sont au chômage en maladie ou en invalidité, leur proportion est de 35% pour les hommes, 45% pour les femmes, selon l'adresse Laurent Berger de la CFDT s'indigne de ne pouvoir discuter de l'allongement de la durée de carrière si on ne résout pas le sort de tous ceux qui sont dehors avant la retraite ces coûts cachés serait de 36 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, sans compter bien sûr les dépenses assurance chômage qui ne sont pas concernés, ici 970 millions supplémentaires pour les arrêts de travail. Vous faites l'impasse sur ces éléments nous manquons des d'une étude d'impact sérieuse pour avoir une bonne vision déséquilibre. Des comptes. D'après les prévisions du COR. Le déficit de l'ordre de 3% et tout à fait résorbable. Résorbable dans les prochaines années, contrairement à ce qu'on nous martèle depuis des mois la pérennité de notre système n'est pas en jeu et ce, même en l'absence de réforme. Le déficit du système de retraite représentent moins de 1% du PIB. Pour rappel, ça a été dit tout à l'heure, la suppression de la AC VAE. 8 5%. Du péage du PIB consacré aux aides aux entreprises le courage se résume à faire payer votre politique en faveur des plus riches sur le dos des plus pauvres. Voilà la réalité. Madame la triche compta. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement pour objet la suppression de l'article qui entérine financièrement la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui veut imposer aux Françaises et aux Français de travailler deux années supplémentaires. Il veut leur prendre 2 années de repos repousser l'âge légal du départ de 62 à 64 ans n'a rien d'inéluctable puisque la trajectoire financière de notre régime et maîtrisé cette mesure causera des inégalités car ce sont les plus modestes, les femmes qui en paieraient le prix fort. C'est un choix de société. Et injuste. Ce report de 2 ans ferme suscite un rejet massif et un mouvement social historique cette grande régression qui plus est imposé de façon brutale dans le cadre d'un véhicule législatif qui ne permet pas un vrai débat en passant par le PLFSS. Le gouvernement recours à l'article 47 ans pour réduire le débat parlementaire. En témoigne le nom d'amendement irrecevables donc au cynisme face aux Français, Emmanuel Macron, ajoute le mépris, la représentation. Nationale. Cette réforme se justifie, dites-vous par le déficit au cours du précédent quinquennat. Les baisses d'impôts au profit des plus riches et des grandes entreprises ont amputé le budget général de l'état de 50 milliards d'euros par an. À cela s'ajoutent les exonérations de cotisations ont tous genres les dernières. Augmenté 3 fois plus vite que les aides sociales et au, au cours de ces 10 dernières années. En 2023, elles représenteront 19 milliards d'euros en partie supporté par la branche vieillesse de notre sécurité sociale, soit un peu plus que les économies que cherche à faire le gouvernement, par cette réforme. Ces exonérations ont un coût pour les finances publiques, ce n'est pas aux travailleurs de le supporter ce déficit qui n'est pas une paille, Monsieur le Ministre, relève d'un choix politique et la dramatisation de ce déficit de votre part relève d'une tromperie. Merci monsieur le président. Mon intervention porte comme pour mes collègues sur la suppression de l'article liminaire et son approche purement comptable. Vous avez insisté tout à l'heure Monsieur le Ministre sur le fait que j'ouvre les guillemets 13 milliards d'euros. Ça n'est quand même pas une paille, fin de citation. Mais je voudrais vous rassurer, Monsieur le Ministre, même à gauche même sur ces bancs, on sait encore faire la différence entre les millions et les milliards. On a tous ici gérer des Budgets dans nos collectivités. Donc on voit à peu près ce que ça peut représenter. Donc nous allons causer recette. Ici, sur ces bancs, nous savons aussi affirmé que le problème n'est pas l'impôt qui n'est pas un gros mot n'est pas la taxe qui n'est pas plus un gros mot, mais la redistribution et c'est bien ça qui fait la différence entre votre approche et la nôtre. C'était d'ailleurs le fondement pour trouver des recettes de la proposition qui a été faite il y a quelques mois d'un référendum d'initiative partagée. Faute de propositions gouvernementales en ce sens sur la taxation des dites des super profits qui selon de calculs aurait pu ramener 10 milliards d'euros dans les caisses, vous voyez que des 10 milliards d'euros au 13 milliards d'euros que vous semblez rechercher. Nous ne sommes pas trop loin et vous M. étant avec certains collègues de la majorité sénatoriale nous dire que le choix des autres pays européens nous oblige, nous qui sommes encore je l'espère une nation souveraine, hé bien nous pourrions faire le même chemin. Pour ce qui est de trouver des recettes en Espagne taxation exceptionnelle prévue pour 23, 2023 et 2024 pour ramener 7 milliards d'euros sur les deux ans et financer divers mesures sociales en Grande Bretagne dont pourront on ne peut pas dire qu'il fasse de la politique gouvernementale avec le couteau entre les dents taxe supplémentaire sur les compagnies nationales exploitant sur le territoire national et compagnie nationale de pétrole avec une taxe additionnelle de 25% qui a également un caractère temporaire, comme c'était notre proposition et en Italie. Je peux en citer d'autres, 10% sur les profits exceptionnels du secteur de l'énergie,

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, la réforme des retraites ne devrait pas passer par une loi de finances rectificative de la Sécurité sociale tant un langage. La vie de toutes les Françaises et de tous les Français et les est inopportune et rejetée par l'immense majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens par toutes les travailleuses et tous les travailleurs du pays dès lors cet article liminaire obligatoire dans une loi de finances de la Sécurité sociale qui entérine financièrement cette réforme des retraites injuste et injustifiée, doit être supprimé. Loin d'être une véritables réformes du fonctionnement global de notre système de retraite cette réforme est purement paramétrique conservatrice injustifiées et injuste. Elle ne répond qu'aux seuls impératifs d'équilibre des comptes publics, à la suite d'une politique intensive de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Fin de la sévère et aux ménages les plus riches. Suppression de l'ISF, création de la flat tax, mais aussi d'un transfert de la dette Covid 19 sur les comptes de la protection sociale. Or, d'autres solutions existent, elles exigent elles exigent de poser la question des recettes du système question absolument taboue taboue pourtant pour votre gouvernement. Pourtant les exonérations de cotisations sociales dont certaines sans aucun effet notable sur notre économie coûteront la branche vieillesse 18 9 milliards d'euros en 2002 soit un peu plus que les 17,7 milliards d'euros que le gouvernement cherche d'ici 2030 à travers sa réforme. D'autant que ces 17,7 milliards et ce comté ne tiennent pas compte des coûts induits du report à 64 ans de l'âge légal du repas. Départ à la retraite pour l'assurance chômage et les minima sociaux, le gouvernement crient à l'urgence. Il est démenti par le conseil d'orientation des retraites par de nombreux économistes par l'intégralité des syndicats et même certaines organisations patronales. Il est urgent de retirer ce texte de reprendre de véritables discussions et d'envisager une véritable réforme qui alliera sauvegarde de la répartition et progrès social.

Je vois le ballet qui est le nôtre, là je suis assis dans mon salon je regarde ce qui se passe au Sénat on voit uniquement la gauche qui se lève et qui défend ses principes et ses convictions. On voit à côté en face. Déjà assoupi d'école. Apparemment, ce serait un peu irrité que nous ferions dans l'obstruction. On a déposé 4335 amendements. Vous en avez écarté milliers. Il en reste 3732, mais malgré cela vous avez l'impression que la componction du responsable qui s'irritent que nous ne débattions pas plus vite et qu'il faut absolument voter, ce qui est le coeur même l'architecture fondamentale du financement sur lequel vous allez vous appuyez-vous dire que les cadeaux fiscaux fiscaux ont été fait forcément ça peut gêner et ça peut irriter. Non, on est dans un exercice absolument dantesque kafkaïen. Je le dis très clairement, j'ai une vingtaine d'années de prestations dans les hémicycles je n'avait pratiquement. Jamais assisté à ça je dois dire effectivement que je n'avais jamais connu l'article 47. 20 jours alors qu'on aurait pu prolonger les débats à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ici même dès qu'on ne n'avait pas touché au dos jours. Aucun jour du Sénat. On aurait pu prolonger le débat et on se satisfait de ça bien sûr, vous avez le droit des, des femmes de votre idéologie votre vision et votre prisme nous aussi nous avons le droit, sans pour autant être taxer qu'on fait dans l'obstruction. C'est un article inique. Nous demandons la suppression de Merci Monsieur le Président. Cet amendement que j'ai déposé aussi de membres de la suppression de certes article liminaire. Particulièrement parce qu'il entérine financièrement une réforme injuste qui ne se justifie que par votre volonté de récupérer des finances sur le travail des Français, et particulièrement sur les plus-préfet Caire et sur les femmes. Elle répond uniquement cette réforme à un impératif de réduction des risques, pas des dépenses publiques mais nous l'avons je pense ici démontré. Il n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme et surtout pas de cette façon et pas avec ce véhicule législatif. Ce n'était pas non plus le moment. Je vous rappelle quand même, Monsieur le Ministre, que les Français viennent de subir la crise sanitaire, la crise économique ils subissent l'inflation les difficultés pour de nombreux français à se à boucler leur budget les difficultés à se soigner à se loger à se déplacer à Sochaux chauffer. Monsieur le Ministre était-ce vraiment le moment de faire cette réforme ne pouvait-on pas attendre de voir les effets de la réforme Touraine. Une autre question pourquoi ne revenez-vous pas sur le ce dogme de non-, renouvellement des fonctionnaires nos services publics ont besoin d'être renforcée, particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la santé et est-ce que c'est pas aussi ce renouvellement ou cette augmentation des fonctionnaires qui permettrait de rééquilibrer un certain ou dans rééquilibrer un petit peu une partie, bien évidemment, c'est vous qui en être. Vous, Annette l'employeur dans c'est vous qui payez les cotisations mais qui devait aussi récupérer les recettes réfléchissez aussi un petit peu donc effectivement vous avez des moyens pour augmenter les recettes des systèmes du système Prenez-les, prenez vos responsabilités. C'est pourquoi ça que nous souhaitons que nous supprimer cet article, que de revenir sur cette réforme des retraites. Merci monsieur le président. Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le dicton populaire mentionne que lorsque l'on veut noyer son chien on dit qu'il a la rage comme le mentionnait tout à l'heure notre collègue Yan Chantrel, cette expression proverbial qui date du XIIIe siècle, époque où il faut le reconnaître, on ne se souciait guère de la condition animale images le fait que l'on trouve toujours une cause afin de se justifier aujourd'hui les déficits de la branche retraite sont présentés comme un épouvantail qui justifieraient cette réforme injuste et qui n'est pas nécessaire. Je ne reviendrai pas sur le rapport du COR que vous bafouez et qui indique que les dépenses sont maîtrisés et qu'il y a certes un manque de recettes et c'est bien sur le volet recettes qu'il faut se pencher. On nous indique également que le ratio actifs cotisants sur retraités se dégrade à terme ce qui est vrai en omettant de mentionner les gains de productivité et la richesse produite par salarié qui elles augmentent plus vite que le ratio lui ne baisse notre système de retraite par répartition doit aussi être un système de répartition de la richesse produite par le travail concernant les incidences de cette réforme sur les autres mécanismes de solidarité, on oublie. Comme l'indique une étude de l'adresse qui s'est penché sur la réforme de 2010, réforme, Fillon, Woerth et qui a reculé de 60 à 62 ans l'âge de la rente traite que mécaniquement les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique, ont vu leur situation se prolonger de 2 ans supplémentaires, générant un surcoût de 600 millions d'euros par an pour ces régimes parce que lorsqu'on est malheureusement au RSA à 60 ans est trop éloignés de l'emploi, on le reste à 62 et on le restera à 64 ans. Le tableau ne tenant pas compte de ces coûts induits. Il est donc naissent. Il est donc un sincère et j'en demande la suppression. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet amendement. Vous imaginez bien, je vous propose de supprimer cet article liminaire, il est en effet hautement symbolique de tout ce qui ne va pas dans ce texte, comme de très nombreux collègues. Je suis très favorable à ce que nous nous attelions à une réforme des retraites à une réforme des retraites mais il faudrait le faire vraiment pas dans ce cadre contraint est tronqué par le que le gouvernement nous impose avec le recours de l'Arctique à l'article 47 tirer hein pas en y consacrant que 12 jours et pas dans le cas d'un PLFSSR. qui limite tellement votre capacité d'amendements et de propositions. Plus de 1000 amendements ont été retoqués avant même que nous puissions discuter certains aurait pourtant permis d'ouvrir des débats positifs comme celui de la reconnaissance de nos responsables associatifs ou par une modification de leur retraite. Nous sommes donc réduits à devoir comme l'entérinent cet article liminaire nous prononcer sur une approche purement paramétrique des retraites mais il n'est pas sérieux d'examiner un texte qui aura de telles conséquences sans même les considérer et pourtant vous avez volontairement écarté les prévisions qu'il en tienne compte. Même les plus sérieuses comme le modèle développé par l'Insee et la direction générale du Trésor dit mésange certes celui-ci démontre les effets négatifs de votre réforme sur le plan macro-économique. Vous avez donc choisi une démarche dite comptable pour ma part je la qualifierais plutôt de cynique. Vous venez en effet simplement chercher de l'argent dans les caisses de retraite fort bien géré par les partenaires sociaux pour compenser, celui que vous n'avez de cesse de jeter par les fenêtre s'cela a commencé avec le quoi qu'il en coûte. Pendant la crise sanitaire et vous avez refusé tout ciblage des aides et encore plus la mise à contribution de ceux à qui la situation profiter cela se poursuit, avec des cadeaux aux plus riches et aux entreprises qui n'ont aucun caractère d'intérêt général. La suppression de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises a été dit tout à l'heure et votre dernière en date, elle coûtera 8 milliards d'euros en année pleine et désormais ce sont les travailleurs qui souvent présenter la facture votre quoi qu'il en coûte, va leur coûter 2 années supplémentaires de leur vie. Revoyez vos prévisions. Revoyez vos priorités et ensuite nous pourrons parler vraiment des retraites d'ici là, je propose la suppression de cet article liminaire basée sur des estimations auxquelles nous ne pouvons faire confiance et sur une démarche trop cynique pour qu'on puisse y adhérer. Merci monsieur le président. Mon amendement est un amendement de suppression de l'article liminaire. Parce que celui-ci entérine financièrement une réforme paramétrique des retraites qui est injuste et qui est injustifiée. Celle-ci répond à un impératif de strict équilibre des comptes publics, à la suite d'une politique extrêmement intensive de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises d'une part par exemple la fin de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais aussi en direction des ménages les plus riches, comme la suppression de l'ISF, la création de la flat tax la flat tax et la liste pourrait être prolongé mais aussi d'un transfert de la dette Covid. Sur les comptes de la protection sociale. Or, d'autres solutions existent bien entendu elles existent, elles exigent pardon de poser la question des recettes du système question absolument taboue pour le gouvernement. Pourtant les exonérations de cotisations sociales dont certaines sont sans aucun aucun effet notable sur notre économie coûteront à la branche vieillesse 18 9 milliards d'euros en 2023, c'est-à-dire sensiblement plus que les 17, 7 milliards que le gouvernement recherche désespérément d'ici 2030 à travers sa réforme. D'autant que ces 17,7 milliards escomptés ne tiennent pas compte des coûts induits du report à 64 ans de l'âge légal du départ à la retraite pour l'assurance chômage et pour les minima sociaux. Monsieur le président. Madame la rapporteure générale nous a bien expliqué hier dans sa DG. Que la modification de ce Plfss, il portait sur 600 millions de dépenses pour les minima de pension et 200 millions d'économies sur le relèvement de l'âge au 1er septembre, ce sont les seules conséquences de la réforme sur le solde de l'année en cours. On est donc en droit de se demander si la brutalité de cette réforme avec application dès le 1er septembre n'est pas là uniquement. Pour justifier une loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Et l'utilisation du 47. Pour mémoire, dès avril 2020 le budget de la Sécurité sociale avait explosé avec plus de 2 milliards pour lambda mais plus de 4 milliards pour la santé publique pour Santé publique France. Et le Sénat n'avaient pas pour autant obtenu un PLFSS. Et notre chiffre. 85 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Le transfert de la dette Covid sur la sécurité sociale, 136 milliards. Et après on va nous raconter que ce sont les retraités qui font le déficit des comptes sociaux. Le déficit des comptes sociaux. Il est parfaitement organisé et je terminerai par une question Monsieur le Ministre tout à l'heure nous a parlé des créations d'emplois. Monsieur le président de la République s'est fait élire sur effectivement un engagement de réduction d'emplois et depuis 5 ans. On entend dire que vous êtes les meilleurs. Alors finalement, est-ce que vous ne nous est-ce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Puisque si tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si la dynamique de l'emploi telle que vous la venter continue. Je ne vois pas où seront les problèmes pour financer les retraites. Merci monsieur le président. C'est ainsi que, mais aussi l'ensemble du texte mérite d'être supprimés. Monsieur le président. Mais mes chers collègues. Ce texte pénalise la majorité des Français les plus fragiles, mais aussi les plus travailleurs, ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui ont été applaudis pendant 2 ans. Ceux qui sont malades avant 62 ans, ce qui ne résiste plus ceux qui sont maltraités, institutionnellement, mais aussi par ses choix. Les choix que vous faites. Messieurs les ministres, les travailleurs identifié sur les emplois nécessaires et utiles. À notre survie pendant la pandémie. Ça rend la victime. Les grandes victimes seront tous ceux, tous ceux qui régulièrement ont été applaudi mais très vite oublié dans votre zone de confort. Vous oubliez ceux qui n'ont pas résisté résisté aussi à la maladie. Ce sont en majorité les femmes. Les femmes des services d'aide à la personne de l'éducation, les caissières, les éboueurs. Ce sont toutes ces personnes qui nous ont aidé à survivre dans notre confort. Et aujourd'hui oubliés et ce sont ces personnes qui seront également pénalisés par ces mesures. C'est injuste. injuste, injustifié. Et à la limite choisirai même que c'est malhonnête de notre part. Je vous remercie.

Le corps le démontre, vous le savez aussi. En revanche, ce dont il s'agit en 1er lieu ici, c'est de la vie de nos compatriotes et de ceux notamment qui travaillent dur longtemps trop souvent jusqu'au soir de leur vie pour faire fonctionner notre économie et nos services publics je pense ici à ceux qui donnent de leur personne et se sacrifie parfois souvent pour que le pays avance malgré tout et on l'a vu, ça vient d'être rappelé avec le Covid. Leur investissement est au fondement du contrat social et nous ne pouvons pas le réduire à une fraction de critères quantitatifs comme le PIB, je le répète Monsieur le Ministre votre approche et partielle partiale économétrie. Incertaine et au bénéfice premier comme souvent de ceux qui ont les faveurs de vos politique depuis 2017. Elle répond aussi l'injonction européenne qui renvoie votre gouvernement et le président de la République à l'état déplorable des comptes de la nation française. Qui sont affectés à la marge par les régimes de retraite et peut-être, en tout cas, je le crois. Et ceux-là sur le seul fondement politiques inavouées par vous parce qu'inavouable aux Français que vous rendez responsable de vos propres turpitudes en matière de gestion et de tenue préoccupante parce que mauvaise des comptes publics. Amartya Sen, le grand économistes disaient que l'économie est une science morale. Il est encore temps pour vous de donner sens à cette parole hein retirant 7 Arctique péri liminaire dont je voterai avec mon groupe, la suppression. Monsieur Marie. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Cet article liminaire entérine de fait une réforme paramétrique injustifiées et injustes. Et particulièrement brutal qui va faire supporter aux travailleuses et aux travailleurs vos choix idéologique. Et votre politique libérale depuis 2017 ou n'avait cessé de réduire les recettes fiscales de l'État. Impôt sur la fortune flat tax CVAE entre autres. Vous n'avez cessé d'accorder des des exonérations de cotisations sociales massives dont 19 milliards sur la branche vieillesse, vous avez mené une politique d'austérité appliquée à la fonction publique qui voit ses effectifs fondre impactant l'équilibre des recettes du régime des retraites et vous avez décidé de transfert de la dette Covid sur la sécurité sociale. Tout cela. PS et vous avez donc décidé de l'impôt sur la vie en privant les salariés de 2 années de retraite souvent les meilleurs quand on sait l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes à 64,4 ans et pour les femmes à 65,9 ans. Vous avez. Décidé cela alors que d'autres solutions sont possibles, mais elles sont tabou pour le gouvernement et pour la majorité sénatoriale. Qu'en est-il de l'égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes qui selon toutes les études permettrait d'engranger 12 milliards d'euros de recettes sur le régime des retraites. Qu'en est-il du taux d'emploi des seniors, le plus faible aujourd'hui en France par rapport à la moyenne européenne. Qu'en est-il du renforcement des services publics. Quand on connaît les besoins de l'hôpital de l'éducation. Qu'en est-il des taxe sur les superprofits, que nous avons proposé qu'en est-il enfin des cotisations sociales sur les revenus hors salaires notamment sur les dividendes. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore Monsieur le Ministre, nous supprimons cet article. Monsieur le président. Messieurs les Ministres, mesdames, messieurs, chers collègues. Cet amendement de suppression concerne l'article liminaire comme de nombreux collègues l'ont déjà expliqué ici. Je voudrais développer quelques arguments. Messieurs les ministres, vous faites bouger uniquement avec cet article liminaire les différents paramètres des différents régimes pour réduire les déficits et trouver les financements nécessaires. Monsieur le Ministre, vous avez fait un choix de facilité. Je pourrais dire même un choix de paresse. Vous avez surtout fait un choix qui est frappée du sceau de l'injustice sociale. Des solutions alternatives exister. Vous auriez pu par exemple lever le pied sur les cadeaux fiscaux faits aux riches et aux très riches. Vous auriez pu aller chercher l'argent où il est. Sur les comptes et les grandes entreprises qui font des bénéfices par centaines de millions et par dizaines de milliards d'euros chaque année. Vous avez préféré pénalisées, les Françaises et les Français. Celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui triment celles et ceux qui souffrent. Mais en faisant cela vous êtes les dignes Ministre des riches et des très riches, comme nous avons un président des riches et des très riches. En faisant cela vous portez un mauvais coup à la justice sociale à la cohésion nationale au pacte républicain. Mais en faisant cela, messieurs les Ministres vous renier l'année l'autre ce que vous défendiez il y a encore quelques mois voire quelques années vous renier toutes les paroles que vous avez prononcé l'année l'autre dans vos fonctions respectives précédente. Il y a quelques années et tout cela, vous comprenez bien que nous ne pouvons pas le tolérer. Au nom de la vérité que nous devons aux Françaises et aux Français, mais surtout au nom de la justice sociale qui nous anime sur ces bancs. sueur. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc dans les préliminaires enfin on commençait à s'ennuyer, voilà qu'on arrive aux préliminaires et je voulais vous dire mes chers collègues. Que j'ai été très frappé au cours des dernières semaines. Par la grande confusion qui régnait parmi les membres du gouvernement. Monsieur le mini j'ai écouté la dernière séance à l'Assemblée nationale sur ce texte. J'ai été extrêmement frappé. Voilà un texte sur lequel le président de la République a décidé de jouer très gros. Il a décidé de s'affronter. À une grande partie du peuple français. Et moi j'avais pensé que dans ce cas-là, il aurait fait très attention à la cohérence des arguments et à la solidité du texte hors jeu. Il reste à ma mémoire cette séance. 1200 euros alors qu'il touche 1200 euros. Monsieur le Ministre de millions de personnes. 40.014 1013 1000 réponses un discours incompréhensible. 17 ans. Alors si c'est ça pour 17 ans. Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont 18 ans 19 ans 16 ans. Un discours que vous avez lu le Monsieur le Ministre, mais vraiment personne n'a rien compris madame qui a pas ce texte est favorable, très favorable aux femmes. Quand on regarde, ligne à ligne. Alinéa après Alinéa on voit qu'ils pénalisent largement les femmes. Alors est-il possible. Monsieur le Ministre de continuer. Alors que nous sommes dans une telle confusion peut être en huit jours avait vu retrouver quelques réponses à ses questions. Mais moi je m'interroge, je considère qu'il n'est pas sérieux. De traiter les choses ainsi. Comme vous l'avez fait jusqu'à présent et je préférerais vraiment qu'on ne parte sur d'autres bases. Monsieur le président. Je vous remercie. Bien je je vois que effectivement le débat avance et que sur cette question. Les arguments les uns et les autres s'enchaînent et viennent. Nous éclairer sur. Sur le sens profond de cette réforme. Je me souviens. Qu'en 2018 puis en 2019, le président de la République a dit textuellement. Reculer l'âge de départ à la retraite. C'est injuste, je ne le ferai pas pour 2 raisons. Pourquoi.

des seniors qui étaient déjà pénalisés parce qu'il n'avait pas de travail pour une grande partie d'entre eux étaient au chômage pourquoi leur infliger 2 ans de plus au chômage. Et il disait, donc ce n'est pas la bonne réforme et proposer une réforme structurelle. Qui a capoté. Depuis on devait discuter d'une réforme sur le marché du travail qui devait nous éclairer. Notamment sur les tendances lourdes et apporter des réponses à ce travail des seniors qui est au coeur de ce que l'on discute, y compris si on doit discuter de la question financière parce que ce n'est pas pareil. Pour les finances publiques. Si des seniors. Peuvent avoir un emploi jusqu'à 62 ans ou si on continue. Ah les cinq 10 dernières années à les laisser de côté et à augmenter. Leur période d'inactivité, jusqu'à 64 ans, ça pèse sur les finances publiques. Et ça vous ne le chiffre est pas alors. Le président de la République avait dit que c'était injuste, il a changé d'avis et nous nous trouvons toujours que c'est injuste, il faut aux plus démunis. Alors que 50 milliards par an ont été dit c'est plus que les entreprises pendant le quinquennat précédent. Merci monsieur le président. Cet article liminaire mes camarades lundi il n'a qu'une seule justification c'est de valider financièrement la réforme des retraites que vous nous présentez les femmes les carrières longues. Les métiers pénibles. Ils sont les grands oubliés de votre réforme. Mais ils ne l'auront de cesse de les défendre le gouvernement Monti ils étaient réforme par le déficit prévu par le corps en 2030 et qui représente 13 milliards et demi d'euros. Oui monsieur Attal. Nous savons ce que c'est 13 milliards et demi d'euros. Effectivement c'est une très grosse somme surtout pour qu'il gagne le SMIC chaque mois mais pour les comptes. Pour le corps, cela représente à peine 3% de ceux qui distribuait chaque année. En aux retraités, c'est-à-dire 345 milliards et le corps est formel, ce déficit est est absorbable et la pérennité du système de retraite n'est pas en danger. La réforme que vous nous présentez donc n'est pas justifiée. En réalité, cette réforme n'a qu'un seul objectif, compenser les baisses d'impôts majoritairement destinés aux grandes entreprises, moins d'un quart a été destiné aux TPE ou PME. Vous nous présentez cette réforme le décalage de l'art de l'âge de la retraite de zones de 64 ans comme la seule solution pour maintenir notre système de retraite. Pourtant d'autres solutions existent, elle nécessite de sortir de votre dogme des baisses d'impôts et de cotisations et de repenser la question des recettes du système, puisque c'est là que le bât blesse. Les exonérations de cotisations sociales coûteront à la branche vieillesse 18 9 milliards en 2023. C'est davantage que les 17 7 milliards d'euros est se par votre four en et ne nous dites pas que ce sont les exonérations comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont permis de créer des emplois. D'abord ce n'est pas vous qui créent les emplois ce sont les entreprises. et puis, ce ne sont pas les agglomérations qui qui ont crée l'emploi, puisque aujourd'hui les économistes disent que les exonérations pour les revenus supérieurs à 1 virgule SMIC n'amène aucune amélioration de l'emploi.

Si Monsieur le. Le président. Cet amendement propose la suppression de l'article liminaire car l'article liminaire finalement c'est le prélude d'un hold-up. Parce que tout ce projet de loi étant hold-up. Hold-up du gouvernement. Pour cacher sa mauvaise gestion. Les plus de 500 milliards de dette construit au cours des 3 dernières années. Les plus de 100 milliards. De dettes qui ont été la dette Covid peut être mais la dette Covid. Qui était une situation politique et qui a été reporté pour plus de 100 milliards sur les comptes de la Sécurité sociale sur seule décision politique. Voilà donc cette situation aujourd'hui. Avec ce projet de loi, vous faites un hold-up sur ce qui constitue le coeur du contrat social français pour masquer votre mauvaise gestion et ça n'est pas acceptable. et. La majorité sénatoriale va se faire complice de cela en ayant. Supprimé déclaré recevable. Des milliers d'amendements qui proposait des sur des sujets de fond comme l'avenir des polypensionnés par exemple sur des sujets qui mériteraient d'être abordée. Nous ne pourrons pas débattre car tous ces sujets ont été déclarées irrecevables je pourrais madame la présidente, je pourrais madame la Sur plusieurs amendements pour montrer à quel point vous voulez escamoter ce débat pour finalement être complice d'un hold-up. Ça n'est pas acceptable, ça n'est Et pourtant si nous devions aujourd'hui, regardez les problèmes de notre pays en face les problèmes de l'Europe en face. Le problème de compétitivité par rapport à la crise de l'énergie. La situation en Ukraine. Est-ce que vraiment nous avons besoin réparer a conclu complice de ce hold-up non. Alors passons aux choses sérieuses et repoussons ce projet de loi. Monsieur le Président Kader. Monsieur le président. Messieurs le Ministre. Je crois qu'il ne vous aura pas échappé que nous ne voulons pas d'article liminaire. Encore quelques-uns à intervenir. En la matière pour essayer de vous en convaincre d'abord bien sûr nos collègues de la majorité sénatoriale. Très simplement, cet article liminaire répond à un impératif qui est celui des de l'équilibre des comptes publics. Faisant état des prévisions les soldes des administrations publiques pour 2023 et c'est là que le bât blesse. Puisqu'en fait vous avez désarmer fiscalement notre pays depuis maintenant 5 ans. allons perdre nous allons perdre 500 milliards d'euros de recettes fiscales et donc la possibilité pour l'État d'intervenir. Et dans ce cadre là dans le CICE. Monsieur Lemoine, c'était 20 milliards d'euros. Je vous rassure. Ces 20 milliards d'euros et ce n'était pas pérenne et c'était pas pérenne et ce n'était pas pérenne. Très simplement, 500 milliards d'euros. Comment vous avez pu ainsi passer un trait de plume sur le sujet. Flat tax créé. ISF supprimé. Exit tax supprimée. Le transfert de plus de 100 milliards effectivement de la dette Covid sur les comptes de la Sécurité sociale. C'est aussi toutes les mesures d'exonération pour les impôts de production et ça fait plus de 30 milliards. Sauf erreur de ma part. Et aujourd'hui et aujourd'hui et aujourd'hui, messieurs les ministres, vous dites aux Français, hé bien écoutez, il y a plus d'argent. Il faut qu'on récupère 17 18 milliards d'euros. Et donc vous allez vous les Français, 18 millions de Français vont payer l'incurie budgétaire qui est la vôtre, Monsieur le Ministre, rappelez-vous de cet adage latin. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous demandons la suppression de l'amendement préliminaire Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est la réforme ou la faillite. Tels sont les propos que monsieur le ministre des Comptes publics non sans elle a prononcé à l'Assemblée nationale. Pour faire accepter votre réforme dont personne n'a encore compris l'intérêt. Le gouvernement aidée par sa béquille droite sénatoriale agite comme un chiffon rouge le potentiel déficit à venir. Quitte à le gonfler artificiellement. J'ai lu dans le dossier de presse qui accompagne la réforme que je cite, si l'on ne fait rien. Le solde du régime des retraites devrait se dégrader. Il manquera 12,4 milliards d'euros en 2027 13, 5 milliards en 2030 et 21,2 milliards en 2035. Il faut dire que parmi les multiples hypothèses que présente le corps dans son dernier rapport. Vous avez choisi celle qui vous arrange. Vous appuyez sur la convention comptable dite équilibre permanent des régimes qui grâce à ce scénario dans lequel l'État diminue très rapidement sa participation au système de retraite. Vous permettez de grossir artificiellement le déficit. Preuve s'il en fallait le corps a détaillé un autre scénario dit effort état constant dans lequel l'État maintient sa participation au régime de ses fonctionnaires. Même si les pensions diminuent. Choisir la convention EPR au lieu du scénario c'est revient à doubler le déficit prévu sur les 25 prochaines années. 05. PIB en moyenne au lieu de sirop de mais ce que, que ce soit 0 5 point de PIB de déficit au 0 2 points. Une chose est certaine. Le système est loin d'être menacé. Je rappelle que les dépenses de retraite s'élève à plus de 350 milliards d'euros chaque année et même si on ne fait rien, la situation ne sera pas hors de contrôle pour autant toute convention et tout scénario du corps confondus le déficit reviendra progressivement à l'équilibre, on faire tripoter sur huit. On est bien loin de la faillite si fièrement claironné. C'est pourquoi je demande le retrait de cet, de cet article liminaire.

Nous le savons tous, la réforme que vous proposez n'est pas une réforme pérenne. Vous dites équilibrer les comptes. Oui, vous allez améliorer à la marge. Les comptes de la Sécurité sociale mais ça n'est pas pérenne car notre système de répartition sera rattrapé par la question démographique cette question démographique d'ailleurs elle n'est pas que française, elle est aussi européenne. Alors comment nos voisins européens et nos partenaires ont-ils répondu à cette épineuse question démographique. Tous sans exception ont créé des systèmes mixtes, qui cumule un système de répartition qui assure une retraite de base. Et un système de capitalisation, un fonds de réserve pour les retraites qui permet au moment du départ en retraite d'apporter un capital qui complètent la retraite, alors ma question elle est très simple, Monsieur le Ministre et ce n'est qu'un amendement d'appel. Pourquoi est-ce que dans ce texte censé équilibrer à terme nos systèmes de retraite. N'avez-vous pas aborder cette question et ne me dites pas que cela ne peut pas se faire à la faveur d'un texte de un projet de loi d'amélioration des finances de la Sécurité sociale a rien ne vous en empêcher. Et vous auriez pu, à l'instar de ce que font les pays européens y compris un grand nombre de pays socialistes et sociaux-démocrates aborder cette question pour apporter une réponse pérenne à l'équilibre de nos systèmes de retraite. Si Monsieur le Président. Moi aussi je vais défendre un amendement de suppression de cet article liminaire blanc pour des raisons quasiment orthogonal. À celle de notre collègue Étienne Blanc qui vient de parler à l'instant c'est pas les mêmes. Raisons parce que justement nous nous déposons cet amendement pour parce que nous voulons conserver un système de répartition juste et favorable aux salariés. Mais je voulais revenir sur la potion que les ministres nous ont présenté tout à l'heure 9 volumes de vinaigre pour un volume de glucose même pas de sirop de glucose pur et vous imaginez que les Français vont absorber cette mauvaise position que vous leur proposez parce que tout votre texte et fait ainsi. Une petite, une petite mesurette par là pour dissimuler le report d'âge et vous nous dites 750 millions pour les hôpitaux, mais comment la gauche ne va pas aller voter les 750 million pour les hôpitaux. Eh bien non, Monsieur le Ministre, nous n'allons pas tomber dans ce petit piège. Nous n'allons pas voter cet article liminaire et je vous mets au défi d'aller dans les hôpitaux, expliquer aux infirmières que la vilaine gauche du Sénat n'a pas voulu voter 750 millions d'euros supplémentaires pour les hôpitaux parce que les infirmières elles savent que votre réforme pour elle elle extrêmement pénalisante, comme l'a été d'ailleurs en 2017 la suppression de 3 critères du compte de pénibilité et en particulier celui des charges lourdes, donc ça ne marchera pas d'aller raconter ça c'est l'enfumage que vous avez choisie comme méthode de communication depuis le début de cette réforme cet enfumage il prend pas les Français vous le montreront le 7 mars encore comme il vous l'ont déjà monté. Montrer à 4 ou 5 reprises et nous ne prendrons pas la mauvaise position que vous nous donnez malgré le mauvais glucose que vous mettez dedans. Merci monsieur le président. Messieurs les ministres, mes chers collègues on amendements identiques, messieurs les ministres, vous voulez redresser les comptes publics et nous sommes d'accord. Monsieur le Ministre, vous voulez sauver la retraite par répartition et nous sommes d'accord. Mais cette réforme qui consiste à repousser. L'âge de départ. D'un trimestre tous les 8 ans. C'est un peu si je peux me permettre le coût de la carte à dépôt différé. Vous savez le banquier il ne retire qu'à la fin du mois. Mais au bout de moins de revenir à la case départ et donc au bout de huit ans, quand on aura prolongé de 2 ans, hé bien on le fera au même point. Alors il faudra, en 2031, passer à 66 ans. En 68 ans à 2039 à 70 ans, 22.047. Où allons-nous nous arrêter. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut explorer d'autres pistes. Effectivement, la démographie, le rapport cotisants cotisés ne permet plus d'équilibrer le régime il faut trouver d'autres recettes. Je proposerai la semaine prochaine à ma demande par exemple de faire contribuer à la sécurité sociale, les cabines de péages autoroutes on a remplacé par l'automatisme. Les salariés qui autrefois en cacher les passagers, je proposerai de taxer les caisses automatiques des supermarchés. Toutes ces entreprises à font des profits non négligeables, ne sont pas délocalisables et pourraient apporter quelques recettes supplémentaires à l'effet de sécurité sociale. Madame hein pour ce. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre a-t-elle nous disiez en préambule de l'examen de cet article liminaire que si nous le suppression. Prions cela empêcherait de payer les fonctionnaires et empêcherait de revaloriser les moyens de l'hôpital public. En résumé, le rejet de cet article liminaire engendré le péril de la France. Ce n'est pas sans rappeler non pas l'excès mais l'outrance du ministre Véran au sortir du conseil des ministres qui a affirmé sans trembler que la journée de blocage du pays du 7 mars, à l'appel de l'intersyndicale ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter l'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe, dit-il écologique agricole sanitaire voire humaine dans quelques mois vous vous situez donc dans le même registre. C'est pourtant un argument Le rejet de l'article liminaire de la loi de programmation des finances publiques, pas de conséquences, le rejet de l'article liminaire ne peut être invoquée comme une épée de Damoclès qui pèserait sur le sort du pays tout entier. Rejetant le largement car le rejeter c'est refuser cette trajectoire austéritaire pour les finances publiques rejetons le car c'est une forme de contestation du passage par un projet de loi de finances pour une réforme des retraites qui devrait faire l'objet d'un projet de loi ordinaire rejetons le car la réforme des retraites que nous discutons n'a pas ou peu d'impact le sur peu d'impact le sur le solde budgétaire de la France cette année, si ce n'est pour ces raisons nous le rejetteront car nous souhaitons rejeté l'ensemble dans la réforme des retraites, ligne à ligne, mot à mot.

Que n'a-t-on attendu entendu pardon sur le rapport du COR. Je voulais un extrait de la page 75 son dernier rapport, le contexte économique qui conditionne la soutenabilité à long terme d'un système de retraite est le reflet de la productivité du travail expression qu'on n'entend jamais du partage de la richesse et des taux d'emploi, fin de citation. Cette assertion démontre que de nombreuses autres facteurs sont à prendre en compte dans nos débats. Telle que la croissance potentielle elles-mêmes calculer précisément à partir de la productivité du travail. L'argument démographique n'explique pas tout, loin s'en faut. Madame, la Première ministre Élisabeth Borne lors de sa conférence de presse de présentation du projet de loi déclaré je cite sans entrer dans des études et des hypothèses complexe il y a une réalité que chacun connaît le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminuent par rapport au nombre des retraités, c'est un fait. Pas un argument politique fin de citation. Comme si, donc il n'y avait pas lieu de débattre c'est factuel. Fermons le banc, l'argument démographique est loin d'être suffisant, on le voit bien, rentrons dans les études au fond de ce sujet le déséquilibre démographique actifs retraités est d'environ 1,7 actif pour un retraité en 2022 contre plus de 4 dans les années 60, ce qui constituerait une impasse certaines pour le régime par répartition. Il faudrait donc travailler plus longtemps dans la vie. CQFD. Argument démographique simpliste il occulte l'idée, s'il y a moins de cotisants par rapport au nombre de retraités, la productivité horaire, c'est-à-dire le PIB par nombre d'heures travaillées a presque triplé, passant de 25 dollars en 1970 à 70 dollars en 2018, le nombre d'heures travaillées 350 heures annuelles depuis 75 due on serait cet argument. selon l'Insee ne tient selon l'Insee, que pour un tiers à la baisse du nombre d'heures travaillées par les salariés à temps complet, restez zen, mes chers collègues. Les 35 heures ne sont pas en cause. Cela aussi c'est un fait et ça n'est pas un argument politique Merci monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le débat porte beaucoup et à juste titre sur la note que votre réforme des retraites va faire payer aux salariés, notamment ceux qui ont des métiers pénibles, aux femmes qui ont des carrières hachées ou à ce qui aurait pu partir en qui aurait pu partir en retraite dans les prochains mois et qui ont l'impression qu'on leur donne 2 ans ferme pour 42 ans de bonne conduite. On évoque moins et je veux le faire à cet instant avec force la note qu'elle va faire payer et peser sur les employeurs publics que sont les hôpitaux et les collectivités. Or, au détour de l'article 6 de ce projet de loi, on apprend que ses employeurs verront leurs cotisations augmenter d'un point quand tu les employeurs privés verront eux leurs augmentations de cotisations, compensée par une diminution de leur contribution à la branche accidents du travail-maladies professionnelles. Selon vos propres estimations, Monsieur le Ministre, ce sont 600 millions d'euros par an entre 2024 et 2028 et 700 millions d'euros à compter de cette date qu', hôpitaux et collectivités devront payer à ce titre, ce nouveau coup dur. S'inscrit dans une longue série de Cuba à l'endroit des collectivités comme la baisse de 0,6% de leurs dépenses en volume inscrite dans cet article liminaire une diminution que mes chers collègues qui siégez sur ces bancs de droite avaient voté notamment dans l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques. Quand nous nous y sommes opposés. Personne ne pouvait dire qu'elle ne savait pas car c'était extrêmement clair. Je vous cite l'article en question les collectivités territoriales, contribue à l'effort de réduction des déficits publics et à la maîtrise des dépenses publiques. Je ne vais pas pouvoir développer sur l'inflation. Les dépenses d'énergies, notamment qui sont extrêmement lourde pour les collectivités aujourd'hui. cette réforme va faire peser davantage encore et ce sera finalement pour nos concitoyens. Une double peine. 2 ans de travail en plus et des services publics en moins. Merci monsieur le président. En fait, pour quelles raisons nous proposez-vous cette réforme des retraites. Telle est la seule question qui vaille, je mets de côté la volonté du président de la République d'apparaître comme un réformateur ou la volonté d'apparaître comme un président qui tient contre la rue qui tient contre le peuple souverain. C'est une marque de fabrique, la fracture de la nation. Quoi qu'il en coûte résultant d'une pratique autoritaire du en même temps, il convient donc d'écouter le président du conseil d'orientation des retraites qui nous dit que les dépenses ne dérape pas mais je cite, elles ne sont pas compatibles avec les objectifs actuels du gouvernement.

dans le programme de stabilité ne sont pas compatibles avec la réduction du déficit public à 2 9 % en 2027. On veut maîtriser voire réduire un peu les prélèvements obligation obligatoire, donc il s'en déduit un objectif sur les dépenses, l'objectif sur les dépenses. Il se formulait de la manière suivante, les dépenses publiques globalement réel de 0 6 %, or vous voyez bien que les dépenses de retraite ne dérape pas, mais qu'elles ne sont pas compatibles avec les objectifs économiques et de finances publiques du gouvernement ce que dit le président du corps comme l'intersyndicale, c'est bien l'incompatibilité du financement du système de protection sociale ici du système des retraites avec la logique austéritaire qui constitue votre projet du gouvernement. Le système des retraites représentent en France 25% des dépenses publiques, soit 347 milliards d'euros. Or le déficit annoncé s'élèverait à 0 7

C'est une hérésie macro-économique, sociale et politique. Je vous remercie monsieur le président. Nous dénonçons le fait que le gouvernement a retenu un mode de compensation pour connaître les projections du sol de système de retraite. En retenant le système dit EPR il avoue qu'il n'entend plus assumer pleinement dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui sa participation au financement des retraites. Notamment à travers les contributions qu'ils versent en tant qu'employeur de la fonction publique d'État, mais aussi en tant que subvention d'équilibre au régimes déficitaires. Or. Si la part des dépenses de l'État. Résulter d'une forme de constance à l'égard du PIB. Nos systèmes serait à l'équilibre aisément à l'équilibre. Le déficit ne dépasserait jamais des 0 4 point du PIB. Soit moins de 10 milliards d'euros constants bien loin donc des 10 milliards. Ah non des Par conséquent. Avec votre dispositif. Nous aurions un déficit qui résulteraient. Plus finalement d'un désengagement par rapport au PIB. Et ceci pèserait considérablement évidemment sur les recettes en matière de recettes en matière de retraite. Au fond, vous créez donc un déficit que vous proposez de combler en demandant aux travailleurs de le faire. Merci de votre attention. Oui nous devons supprimer cet article liminaire parce que nous avons dans ce débat, un gros problème de vérité, de sincérité avec les chiffres. Vous nous dites que cet article il présente en quelque sorte les perspectives d'équilibre du système en fait en vérité cet article ils consacrent un sous-financement organisé et programmé du système par répartition et vous le faites pour ouvrir la voie par paliers à la capitalisation. Le président Larché interrogé dans Le Figaro hier, aujourd'hui je sais. Oui oui enfin ces jours-ci dit sur la capitalisation. Ça n'est pas la question du moment du moment. Sauf que dans le même journal 44 parlementaires de droite viennent de signer une tribune qui s'appelle osons la retraite par répartition. Par capitalisation. Or il y a quand même du beau monde dans ce projet dans ce de cette tribune, monsieur Karoutchi, 1er vice-président Madame Primas, président de la commission économique Madame Gruny vice-présidente du Sénat Madame Delattre vice-présidente du Sénat, monsieur Longeot, président de la commission du développement durable. Donc ça ne sont pas des frondeurs qui signent cette tribune, c'est le coeur de la majorité sénatoriale. Et dans cette tribune, vous nous dites, vous nous dites. La retraite par capitalisation. Quoi qu'il arrive, sera le point cardinal de la prochaine réforme de notre système de retraite. Donc, c'est bien cela que vous visez. Et c'est pour ça que vous allez voter dès demain ce projet en nous disant nous sommes là pour sauver la retraite par répartition. En vérité vous préparer la mort de ce système et le gouvernement le sait pertinemment, et c'est pour ça que cet article liminaire est un article mensonger sur les objectifs véritables de cette réforme.

Qui est brandi en totem par les partisans du toujours moins d'impôts, alors je vous pose la question, est-ce que tous les travailleurs et les travailleuses qui vont se taper 2 années de plus de travail vont pas payer d'impôts. Vous avez la réponse. Ils vont payer des impôts. Et c'est d'ailleurs dans vos éléments de langage. J'ai compris qu'il avait 3 possibilités pour financer la retraite vous me dites si je me trompe, messieurs les Ministres baisser les pensions de retraite on l'enlève. Travailler plus longtemps et 3ème argument augmenter les impôts donc les prélèvements obligatoires sur les deux premiers arguments, on va se focaliser sur le 3ème. Le taux de prélèvements obligatoires est annoncé à 44 9 points de PIB. Et. Franchement il faut se dire les choses. Depuis 1965, le PIB est en baisse. Donc il y a plusieurs responsabilités politiques, y compris la votre maintenant mais celle de gouvernements antérieurs. Les prélèvements obligatoires, ils augmentent en proportion du PIB parce que celui-ci ne croit pas croît moins vite, c'est pour ça qu'on a les chiffre qu'on a là et en 2021, le solde de prélèvements obligatoires est environ de 4 pont au-dessus de la moyenne de la zone euro c'est les comparaisons vous nous faites régulièrement. Mais ce que vous dites pas, c'est que les protections sociales sont 5 points supérieur donc qu'est-ce qui se passe dans notre modèle français y compris et que ce débat sur les retraites, c'est que nous on prélève plus, c'est vrai. Mais on redistribue plus et ce ruissellement là les Français et les Françaises et notamment les plus modestes en ont besoin parce que c'est quoi, c'est pas de l'argent qui s'évapore dans les administrations publiques et qui quitte le circuit économique, vous savez ce que c'est, c'est nos cotisations sociales dont 1,3 points sont. Nos prestations sociales qui sont 5 fois supérieurs. Voilà la réalité des chiffres du modèle social français et c'est ce qui nous permet d'avoir une république unitaire qui est une République qui est solidaire. Voilà et c'est votre projet de réforme et notamment cet article liminaire, qu'il le met en cause et il faut dire la vérité je finirai Monsieur le Président. Les impôts sur la consommation des ménages. Je le dis à tous mes collègues. Il rapporte 4 fois plus que l'imposition sur les bénéfices des sociétés. Vous trouvez ça normal qu'on vous trouvez ça juste. Alors on va demander l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements qui ont fait l'objet d'une discussion commune et qui ont la particularité d'être totalement identiques. Madame l'arbre. Merci monsieur le président. Messieurs les Ministres, chers collègues, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Alors je dois dire que finalement cet article liminaire, il a servi de tribune à chacun d'entre vous. J'ai eu le sentiment d'assister à la 3ème discussion générale parce qu'on a eu un petit peu de tout mais est-ce que ça nous privera encore d'expression, je ne le pense pas Nous allons savourer à certains dire disent qu'ils vont voter demain mais bon ça c'est c'est peu prévisible. Je voudrais commencer par dire que. Cet article liminaire, en fait, il est obligatoire, donc vous parlez tous de le supprimer, mais en fait, ça date déjà de la loi de 2001, la loi organique des des des lois de finances la LOLF. Donc, il est obligatoire et qu'est-ce qu'il nous donne cet article il nous donne en fait les prévisions de solde structurel et de soldes. Effectif. Moi j'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Dans dans vos propos. qu'on, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet article en fait que. Le seul de public, de l'ensemble des administrations publiques retenu pour 2023 s'établit à moins 5% du PIB. Donc ça c'est intéressant de connaître ce chiffre et il faut le retenir. Je pense que vous avez aussi noté qu'il est assez semblable finalement au tableau des prévisions de la loi de financement de 2023 donc. On peut dire effectivement que cette loi. Sur les retraites n'aura pas beaucoup d'incidence mais tout de même, il s'est passé des choses au cours de ces de ces quelques mois qui ont fait que quelques points ont varié. Je ne vais pas vous les donner, moi je me suis arrêté surtout au tableau des soldes, recettes et dépenses. Des administrations de Sécurité Sociale parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Et et et je regarde la décomposition de ce tableau. Et je vois que par exemple quelles observations. Nous pouvons faire d'abord qu'il y a un excédent de 21,1 milliards d'euros et là je voudrais me tourner vers mon collègue Pascal Salvodelli parce que tout à l'heure, il disait mais finalement en quelques temps on peut on peut rattraper. Le déficit mais en réalité, c'est 21,1 milliards d'euros proviennent essentiellement de l'amortissement de la dette sociale. Qui. Procède de la. Et là on a un montant de 16 4 milliards d'euros qui finance justement ces 21 milliards d'euros dont je parlais En réalité, Monsieur Salvodelli, on va pas résorber la dette comme ça parce qu'on a déjà encore 155 milliards de d'être. Qui ne sont pas amortis. Donc je vous demande un petit peu d'attention et un petit peu d'économie. Et je voudrais aussi vous dire que. La situation est favorable sur l'assurance chômage et ça c'est un indice important parce qu'on vient de vivre 2 années successives Qui ont été compliquées avec la Covid, avec le temps partiel et ça vraiment été. Difficile pour l'Unédic et donc là on est sur une dette. Qui a atteint donc plus de 63 milliards d'euros. Justement, après ces années difficiles et là on aura finalement une dette qui qui va décroître jusqu'à 55 milliards d'euros pour 2023 donc c'est mieux donc on observe quand même des des des avancées significatives. On pourrait parler aussi des régimes de retraites complémentaires où là effectivement il y a aussi des aspects positifs. Donc. En 2023, la situation est est moins favorable mais il y a aussi une prise en compte des effets en année pleine des majorations de pensions et une décélération attendue de la croissance de la masse salariale. Ce que je, je voudrais dire aussi c'est qu'il y a dans ce tableau, le fait que. Un amendement a été voté à l'Assemblée nationale qui donc. Rajoute 750 millions d'euros sur l'Ondam donc ça ça a pas pu être intégré à l'article 15 puisque c'est l'article 15 qui consacre en quelque sorte cette augmentation pour l'Ondam puisque l'Assemblée nationale n'a pas été au bout de de ces travaux. Moi je voulais simplement dire quelque chose parce que il y en a qui ont parlé et on aura sans doute l'occasion d'en parler des cotisations quand on on on on regarde quel est le pays qui a le plus de charges sociales au monde. Hé bien vous trouverez. C'est très facile, c'est la France sur un bulletin de salaire sur la un bulletin de salaire, hé bien c'est 62% de charges sur un salaire brut par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et si on augmente encore plus. Et je peux vous dire que les salariés, eux ils le savent ça parce que ça fait aussi une part de moins sur leur leur leur nette et je voudrais aussi vous dire que quel est le pays le plus généreux au monde quand vous tapez aussi sur Internet hé bien c'est la France. Donc je crois qu'il faut arrêter de pleurer. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. merci Monsieur le le président a effectivement beaucoup de sujets ont été abordés à l'occasion de ces amendements de suppression sur l'article liminaire, j'avais déjà répondu sur l'article liminaire au moment de la discussion sur l'article et je remercie le rapporteur général qui a très précisément évoqué les tableaux de chiffres je m'arrêterai donc sur un certain nombre d'arguments qui ont été relayées par mesdames et messieurs les sénateurs. Je veux redire que sur la question du déficit Madame Briquet est notamment revenu sur le sujet en disant effectivement qu'il pourrait être pire. Mais la réalité c'est qu'il serait pire quoi. Si nous n'avions pas créer 1.500.000 emplois depuis 5 ans et c'est grâce. Notamment à la politique qui a été menée par la majorité et le gouvernement parce que les entreprises créent des emplois, mais il faut qu'elle puisse créer des emplois et pour ça il faut que le coût du travail baisse et il a baissé parce qu'on a fait on a pris des mesures. Et la 2ème chose et la 2ème chose c'est que si le déficit n'est pas plus important, c'est aussi parce qu'il y a eu la réforme Woerth en 2010 et la réforme Touraine en 2014. S'il y avait pas eu la réforme en 2010 d'Éric Woerth. La réforme de Marisol Touraine, en 2014 on aurait un déficit beaucoup plus important et dans quelques années quand certains aborderont la question du déficit et diront, il pourrait être pire ils diront, heureusement qu'il y a eu la loi du soft en 2023 pour nous empêcher d'avoir un déficit plus important bien sûr, bien sûr et d'ailleurs les majorités qui se sont succédé ne sont pas revenus sur les réformes précédentes, il y a eu des adaptations et c'est normal, notamment en 2012 à l'arrivée de François Hollande pour les carrières longues pour les 60 ans, mais la majorité de l'époque n'est pas revenu sur les 62 ans. Serait grand. Mais non ben non désolée c'est c'est je n'ai pas encore engagé comme je suis aujourd'hui. 2ème, chose que je voulais dire. D'abord. Vous avez abordé. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. C'était monsieur Kanner notamment Madame Briquet aussi et d'autres sur la question de ce que vous avez appelée des cadeaux fiscaux des pertes de recettes. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le déficit des retraites. Pourquoi. Alors que. Mais nous on ne crie pas quand vous vous intervenez avec Olivier Dussopt, donc laissez-moi, laissez-moi parler. Bah oui mais un peu de réciprocité. Suivez. On a d'abord effectivement il y a eu des baisses de cotisations sociales, elles ont été. À la Sécurité sociale par le budget de l'État. Donc les baisses de cotisations. Sont compensées par le budget de l'État. Première chose 2ème chose. 2ème chose comme le travail coûte moins cher parce que les cotisations baissent il y a plus de personnes qui travaillent, 1.500.000 emplois créés. Et donc des recettes en plus de cotisations sociales pour notre sécurité sociale, 25 milliards de cotisations sociales payées en plus depuis 5 ans parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, parce qu'on a baissé la pression fiscale sur les entreprises. Première chose 2ème chose on collecte plus de recettes fiscales depuis qu'on a baissé les impôts sur l'activité économique et des entreprises. Je vous donne un exemple, l'impôt sur les sociétés. Il était à 33%, quand Emmanuel Macron a été élu, on l'a baissé à 25%. On reçoit, on perçoit plus d'impôt sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. Pourquoi parce que ça rapporte plus de taxer moins un gâteau qui grossit que de taxer plus un gâteau qui rétrécit parce que vous le surtaxer. C'est de la pure logique et c'est de la logique qu'on voit aujourd'hui à l'oeuvre dans notre monde économique parce que plus on baisse les impôts plus l'activité économique se déploie et donc plus on perçoit de recettes fiscales pour nos politiques publiques et et donc oui, je vous confirme, je vous confirme Monsieur Savoldelli qu'on a toujours le 2ème. Taux de prélèvements obligatoires sur les 38 pays de l'OCDE. Malgré toutes ces baisses d'impôts. Vous considérez que c'est une médaille d'argent qu'on devrait avoir la médaille d'or. Nous, nous considérons. Que c'est quand même bien d'essayer de revenir dans la moyenne des pays européens. Parce que quand une entreprise ou. Un investisseur se pose la question de, est-ce qu'il veut implanter son activité qui compare de pays, la France et l'Allemagne par exemple qui votent les impôts de production sont 4 fois plus élevé en France qu'en Allemagne. Ben il va plutôt choisir d'aller en Allemagne qu'en France, c'est pour ça qu'on baisse les impôts de production, c'est ça la réalité. Je veux enfin revenir sur l'intervention de monsieur Valeix. Vous avez abordé la question des superprofits. Moi je veux rappeler que nous avons mis en place et on se souvient de la longue soirée que nous avions eu sur un amendement très très long, avec beaucoup de sous-amendements une taxation des superprofits des énergéticiens dans le PLF 2023. Estimé alors à 11 milliards d'euros. Donc on a fait cette taxe mais je veux juste dire que moi je suis très sceptique, si ce n'est inquiet de l'idée qui est véhiculé de lier notre système de retraite à une taxation des superprofits. Si vous dites que le financement de notre système de retraite doit dépendre d'une taxation des superprofits. Qu'est-ce qui se passe les années où il y a pas de super-profits ben on baisse les retraites et on dit désolé mesdames et messieurs les retraités, il y a pas eu de profits cette année donc on est obligé de baisser leurs retraites. C'est ça le système dans lequel vous voulez mettre nos retraites. Ça serait dangereux pour nos retraités enfin. Je veux le dire et je pense que vous le savez ça d'ailleurs c'est pour ça que les amendements que vous proposez. Il propose pas de taxe étant les super profits que de taxer les Français qui travaillent. C'est ça la réalité. Alors tout à l'heure on m'a dit tout à l'heure on m'a dit faut pas citer l'Assemblée nationale. On est ici au Sénat, donc je vais citer le Sénat et les amendements que vous avez déposé. Amendement 28 57 donc du groupe socialiste proposé de créer un forfait social à 20% sur l'intéressement et la participation. Il y a 5 millions de salariés qui reçoivent de l'intéressement et la participation. Ça veut dire très concrètement qu'il y en a même plus que 5 millions, ça veut dire très concrètement vous dites aux millions de salariés aujourd'hui en France qui reçoivent des primes d'intéressement ou de participation du partage de la valeur que vous allez les taxer à 20%. Aujourd'hui vous avez sur une prime d'intéressement de 1500 euros si on applique votre taxe à 20%. Ça veut dire que le salarié qui devait recevoir une prime d'intéressement à 1500 euros ben il recevra que 1200 euros. Excusez-moi, ça s'appelle pas les super profits, ça s'appelle les salariés qui travaillent 2ème chose amendement 26 28 toujours, le groupe socialiste, vous augmentez les cotisations vieillesse des entreprises. Non mais ça a l'air de vous déranger que je je mette à jour ce que vous avez parlé de tout. Vous avez parlé de tout sauf des amendements de suppression et moi j'ai pas le droit de parler des amendements de création de taxes. Ce que vous faites. Amendement 26 28 proposé d'augmenter les cotisations vieillesse des entreprises ça veut dire que pour nos artisans nos commerçants. Vous leur dites. Nous proposons d'augmenter vos cotisations et donc ça coûte 400 au 440 euros de plus par salarié a recruté amendement 28 55 toujours, le groupe socialiste. Celui-là je pense que c'est le plus dur, enfin le plus difficile. Vous revoyez complètement le système de la CSG en créant des nouveaux taux de CSG. Et donc je vais vous donner un exemple, vous créez un taux de CSG à 7,5% pour un revenu fiscal de référence entre 19.200 euros et 29.800 euros. Aujourd'hui un retraité qui gagne 1600 euros. Son taux de CSG c'est 6,6% avec votre amendement. Son taux de CSG passe de 6,6% à 7,5%. pour pour porter un amendement qui dit à tous les retraités qui ont 1600 euros de retraite, on va vous prendre 173 euros de pension que vous aurez en moins. J'appelle pas ça les superprofits non plus. Oui. Amendement c'est l'amendement 28 55 il est consultable par tout le monde.

de pouvoir d'achat. Je continue puisque vous avez l'air gêné que j'ai, alors je ne sais pas non plus la réalité quoi votre projet politique. Amendement 25 28 Monsieur Gontard. Vous avez l'air de pas être content mais je vais le citer. Vous supprimez les allégements de cotisations sur les bas salaires. Ça fait une augmentation de 39 milliards d'euros de cotisations pour les entreprises, c'est l'amendement 25 28 là aussi est consultable. Donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que pour un salarié au SMIC ça coûte aujourd'hui à l'employeur. 1780 euros de le payer. Vous le passer à 2500 euros pour l'employeur dans plus 700 euros ça veut dire qu'un boulanger, un artisan, un commerçant qui a trois salariés au SMIC, vous lui dites qu'il faut que vous en licenciez hein pour payer les charges supplémentaires qu'on vous demande pour les deux autres j'appelle pas ça les superprofits non plus. je termine et c'est c'est le dernier, je vous rassure, je termine avec l'amendement CRCE parce que vous auriez été déçue que je ne vous cite pas. L'amendement 42 67. Vous augmentez les cotisations patronales et salariales et salariales Ça veut dire qu'avec cet amendement qui augmente d'1,9 points les cotisations salariales pour tous les Français qui travaillent. Un ouvrier qui gagne 1800 euros par mois. Vous prenez 525 euros de pouvoir d'achat. Alors pour conclure, je dirais que quand j'entends monsieur le comte nous parler de hold-up. Quand j'entends Madame Rossignol nous parler de potion amère. C'est plutôt un hold-up et une potion amère pour la classe moyenne, qui travaillent dans notre pays que vous proposez pour financer les retraites, ça n'est pas notre projet politique.

tout à l'heure, il se plaignait un peu d'être seul dans cette avalanche d'amendements de ce côté de l'hémicycle mais je vais lui dire que je veux le remercier, parce que son amendement très utile dans le débat est très éclairant, Pierre Laurent, a expliqué le la tribune dans Le Figaro effectivement où certains appellent de leurs voeux une marche progressive vers la capitalisation et on sait ce qu'il en coûte. Et je voudrais donc d'abord ça montre bien, on comprend la genèse de l'Accord fondamental entre le gouvernement et la majorité sénatoriale. Tout cela est très respectable mais contestable. Et notre collègue a dit que tous les pays européens se sont orientés vers cette option. Je voudrais évoquer le cas de la Suède. Il y a 20 ans, ils ont mis en place une réforme de leur système de retraite comme nous le faisons ici ils ont repoussé l'âge à 65 ans et ils ont introduit un système par capitalisation. le responsable de la Sécurité sociale suédoise à l'époque un certain monsieur Karl Gustaf Scherman. Était-il initiateur du projet et ils ont fait le constat, quelques années plus tard que les pensions des retraités suédois ont PC. Une étude de la caisse des pensions réalisé il y a 3 ans. A établi que 72% des hommes et 92% des femmes ont subi une baisse de leur pension et de leur pouvoir d'achat. Conclusion de monsieur Karl Gustaf Scherman ne recopier pas le modèle suédois, aurait-il dit à monsieur Macron président de la République française au retour de la tournée africaine je suggérerais monsieur Macron d'appeler Stockholm pour savoir ce qu'il en est. Souvenez-vous, souvenez-vous Monsieur collègues. Du scandale Enron aux États-Unis il y a 21 22 jan là les fonds de pension c'est vers c'est vers ça qu'on veut aller et il y a quelques semaines au Royaume-Uni il y a eu aussi fin septembre. Les fonds de pension britanniques ont frôlé la banqueroute après une panique sur les marchés financiers ces géants, chargé de l'épargne retraite des habitants avaient misé sur la spéculation. Si c'est ça qu'on veut. Vous ne trouverez en face de vous, merci. Madame par pour expliquer son vote. Merci monsieur le président. Alors oui bien sûr, nous savons que l'article liminaire est obligatoire et donc si nous voulons ces suppressions c'est bien justement parce que nous ne sommes pas d'accord. Avec la loi de finances 2 rectificatif de la Sécurité sociale mais je voudrais répondre à tout ce que j'ai entendu. Il paraît qu'en allant sur internet, j'ai découvert un on voit qu'on est le pays, il est le plus généreux. Eh bien oui, mais nous, nous nous félicitons d'être un pays généreux. Nous nous félicitons d'être ce pays qui a permis à ce que les enfants ne travaille plus. Il y a fort longtemps dans les mines à ce que les gamins aillent à l'école jusqu'à 16 ans. Oui, oui, ça vous fait rire ou ça vous fait rire, mais enfin c'est toute l'histoire de notre protection sociale à ce qu'une retraite ait été créée à ce que l'hôpital public existe, oui nous en sommes fiers, nous n'allons pas nous en excuser et notre rôle aujourd'hui tiens à ce que on ne personne ne puisse toucher à ce niveau de protection sociale. Vous dites que. Nous devons baisser les cotisations sociales. Mais alors est-ce que vous assumez qu'en baissant les cotisations sociales, on baisse le niveau de prestations. Est-ce que vous l'assumer devant les Français, finalement est-ce que vous êtes en train de dire aux salariés de ce pays, nous allons baisser votre niveau de protection sociale et ce qu'ils pourront continuer à être protégé au maximum, hé bien ça sera ceux qui seront capables de se protéger eux-mêmes par leur propre richesse personnelle. Est-ce que c'est ça que vous allez dire aux Français et enfin pour terminer. Monsieur le Ministre, fait beaucoup de comparaisons. Moi je voudrais rappeler qu'en 2012. Nous sortions même pas encore tout à fait des des de la crise financière liée aux subprimes. Je voudrais aussi rappeler que nous étions au tout début du fameux papy boom. Et aujourd'hui nous nous allons commencer à en sortir, donc il faut comparer ce qui est comparable. Et je terminerai en disant que vous parlez des boulangers, occupez-vous de leur facture d'électricité avant toute chose. Oui monsieur. Le le le ministre Atal vous répondez sur des amendements que qui ne sont pas concernés par. par cet article, on aura tout l'occasion de vous expliquer parce que vous comprenez pas bien les choses entre justement aider les plus démunis et taxer les plus riches effectivement parce que vous les avez bien aider tout au long de ces dernières années, alors qu'ils n'en n'ont vraiment pas besoin mais nous aurons tout l'occasion de nous expliquer là-dessus mais par contre il vous avez pas répondu sur toutes les interventions. Pourtant il y en a eu quelques-unes. Concernant l'article liminaire ça j'aurais bien aimé vous entendre d'ailleurs. Si jamais vous vous, vous ne le saviez peut-être pas, je vais vous apporter une petite information cet article liminaire justement il se fonde sur un projet de loi qui n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale elles-mêmes. Le 1er alinéa de l'Arctique mentionne en effet les prévisions de ces mêmes agrégat tels que figure dans le projet de loi de programmation des finances publiques publiques pour les années 2023 2027. Le gouvernement présente donc un texte fondé sur un projet de loi que le Parlement a rejeté. Comment est-ce possible. Donc nous on demande justement la, la, la suppression à travers tous nos amendements qui visent à à dénoncer quelque part. Cette gabegie je dirais l'Arctique présente une hausse de 400 millions d'euros de la branche vieillesse qui correspond à des mesures d'accompagnement, issue de la présente loi, notamment la question du minimum contributif ou encore des éléments de l'article 9 relatif à la pénibilité. Or ni ni nous n'y voyons pas les baisses de dépenses ni les hausses de recettes qui seraient générés par les mesures d'âge censée entrer en vigueur à partir du mois de septembre prochain. Où sont les économies. Vous n'y avait pas répondu. Comment pouvez-vous affirmer que cet article est sincère. Alors que les économies générées par l'accélération de l'entrée en vigueur de la mesure d'âge à partir de septembre prochain ne figure pas dans le texte. C'est ce que nous aimerions savoir et c'est pourquoi nous avons de déposer ses amendements de suppression afin de dénoncer l'inceste l'insincérité du texte et ses mensonges. Merci monsieur le. Le président tout d'abord je voudrais remercier le notre ministre des Comptes publics parce que si à, à chaque fois que vous devez donner l'avis du gouvernement. Faut tout donner l'avis du gouvernement sur toute une liasse d'amendements, nous n'avons pas fini de débattre donc merci. Deuxièmement, madame la rapporteure. Lorsque vous dites. Finalement, nous sommes le pays. Qui ont qui a les charges sociales les plus élevées d'abord charge non cotisations et deuxièmement c'est totalement inexact. Voyez vous j'ai été employeur en Pologne. Hé ben les taux sont supérieurs. Bien évidemment, parce que lorsque les salaires et malheureusement ils sont nombreux, ils sont inférieurs à un viol de 5 SMIC les cotisations ne sont pas si élevé que cela. Ça a relevé d'une politique économique pendant longtemps à des moments où effectivement il fallait peut-être. Faire en sorte. D'avoir une politique dynamique pour résorber le chômage aujourd'hui, j'entends plus tôt que nous sommes dans une période de tension sur le marché du travail, donc à partir de là la priorité ça devrait être d'augmenter les salaires. Pas d'augmenter les primes comme ce que vous nous avez fait pendant, c'était l'été dernier. Parce que lorsqu'on ne, on augmente les primes. Il y a pas de recette sociales en plus. Et c'est votre politique de primes de multiplication des primes plutôt que de d'augmentation des salaires qui affaiblit aussi les comptes sociaux. Monsieur le Ministre, si vous voulez rétablir maître rétablir donner plus de moyens pour la sécurité sociale, il faut augmenter les salaires, ça mettra ça fera rentrer des cotisations et deuxièmement. Il n'est pas exact. Malheureusement. De dire que les retraites vont peser de plus en plus dans le PIB, parce qu'il faut pas simplement face ça fait 30 ans qu'on nous raconte regardé la démographie et et c'est juste intenable. Regardez les chiffres, pas de cette manière là comme ça au doigt mouillé mais regardez les chiffre ce que ça pèse dans le PIB. Regardez les chiffres du corps. Oui ça a augmenté entre 2000 et 2020 mais aujourd'hui c'est stable et ça va baisser. Et cette baisse elle devrait nous inquiéter, parce que cette baisse il faut conclure baisse elle devrait vous avez laissé votre temps seulement, elle devrait nous inquiéter. On nous avons.

Pour lui dire que la capitalisation, ce n'est pas une cagnotte, ce que vous mettez sous votre lit, qui ne prendrait pas donc sur les dépenses du PIB. Non c'est une part de PIB quand il faut la la dépenser pareil donc c'est une île. Oui une illusion. Je ne dis pas une ineptie économique car in fine et répartition ou ou capitalisation les pensions sont toujours prises sur le PIB bé réel. Donc la différence n'est pas dans les, dans la part de du PIB effectivement c'est la différence c'est entre une solidarité redistributive ou l'assurance selon ses moyens seulement. Vous savez messieurs les les ministres il lui, il a fallu beaucoup d'interventions à l'Assemblée nationale pour lever le mensonge sur les minima contributif. J'interviendrai autant de fois qu'il le faudra pour vous faire admettent. Que le maintien de la situation de départ à 62 ans des invalides n'est pas un surcoût de la réforme. Ce n'est pas une économie. Certes vous baissez pas les pensions, mais ce n'est pas non plus un surcoût c'est neutre donc en le mettant comme surcoût. C'est un mensonge. Je vous demande donc officiellement de le sortir des mesures financières, ce qui nous ramène les mesures dites sociales à 3 milliards, soit un 6ème des gains que vous prenez sur les travailleurs et d'admettre que le solde du coup n'est pas de 0 mais d'un excédent de 3 milliards, trois milliards pour

Oui, mes chers collègues. Bien sûr je voterai cette. Ce retrait de de l'article liminaire. J'ai déjà expliqué comment vous aviez gonflé. Femme. Gonfler le déficit en sous-, estimant les recettes. J'aurais pu prendre un autre exemple qui est le taux d'activité des femmes qui dans vos simulations ne doit pas bouger. on aura toujours de grandes inégalités sur l'accès au travail des femmes, je ne parle même pas des salaires dont chacun sait que s'ils étaient à égalité les caisses de retraite seraient quasi équilibré. Je veux en effet et je reprendrai pas les arguments sur les impôts. Que tous les collègues de gauche ont défini, on décrit tout à fait parfaitement. Je vous dites Monsieur le Ministre, que nous serions pas attentif aux aux Français moyen. Cadeau salarié moyen. Je vais vous lire les propositions de la CFE-CGC. Dont chacun notre vous voit bien que c'est pas des gauchistes bolchévique. Irresponsable. Quant à la gestion. il constate. Que la part dans le PIB de la valeur ajoutée a tellement basculer. Du monde salarié. Vers le capital qu'en effet, à partir du moment où les salaires. Et là tout ce qu'a dit monsieur le comte sur les prix, mais juste à partir du moment où les salaires n'augmentent pas. Vous pouvez toujours parler du déséquilibre entre les actifs de d'actifs. La réalité c'est les masses salariales.

Et que par contre, la part revenant aux actionnaires est passé de 5 2 à 15. 8. Ont très peu d'années. Alors il y a de la marge pour équilibrer tout ça.

Monsieur le président. Messieurs les Ministres. Je suis surpris d'avoir entendu de la part du ministre Atal tant de. Propos et de réponses à des amendements qui n'ont pas été débattu par contre je suis déçu de ne toujours pas avoir entendu la réponse à la question que je posais pourquoi cachez-vous aux citoyens et aux parlementaires la note d'analyse du Conseil d'État qui montre que vous choisissez un véhicule inapproprié à cette réforme. Donc je le redis, j'attends des ministres plutôt des réponses à ces questions je dis aussi quand vous lisez les sondages sur l'appréciation de cette réforme de des retraites. Messieurs les Ministres ayez conscience que vous êtes en train de mettre un pays sens dessus dessous. Regardez que même chez les sympathisants les républicains, 58% se disent défavorables à cette réforme, surtout les rangs de ce pays, les gens vous disent, retirer cette réforme alors commencer par la transparence. Respecter chercher d'autres solutions. Le développement des salaires l'augmentation des salaires. L'augmentation du travail des femmes et n'allait pas chercher à voler 2 années de vie de nos concitoyens. Ces deux années. Vous me disiez monsieur Dussopt. Il suffirait de presque rien hier après-midi oui. Il suffirait de presque rien ne pas voler 2 ans aux Français. Si le président Laurent. Oui, je voudrais dire à monsieur le ministre est à madame la rapporteure puisqu'on va passer 10 jours ensemble. Il vaudrait mieux s'entendent sur le sens des mots dans cette discussion. Des mots qu'on va souvent entendre. Alors tout le monde ici est soi-disant pour la répartition mais tout le monde les même pas tout le monde mais en tout cas à droite et au banc du gouvernement est très inquiet des cotisations des impôts mais un système par répartition, c'est quoi. Ce sont des cotisations prélevées sur la valeur ajoutée du travail créées par le travail pour financer les retraites, l'assurance maladie s'il n'y a pas de cotisations sociales. Il y a pas de système par répartition, c'est le principe même de ce système, on prélève directement sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise par le travail par le travail des salariés pour financer ça. Et ce ne sont pas des charges madame la rapporteure. La retraite, ça n'est pas une charge, c'est une libération après une vie de travail, l'assurance maladie. Ça n'est pas une charge, c'est ce qui nous a sauvés pendant la pandémie. Le travail c'est la richesse créée qui va permettre de tout financer, donc vous ne pouvez pas en permanence nous dire, nous sommes pour le système par répartition et en permanence nous a expliqué que le problème c'est ce qui finance le système par répartition, il faut que nous vous assumiez les choix, si vous êtes pour un système par répartition. Alors il faut près de protéger la cotisation sociale et il faut même oui nous l'assumons la développer. Si les besoins sociaux le mérite et le pays sans sentiras mieux ça fera aussi du développement économique. C'est d'ailleurs le compromis qui a été passé entre un communiste embrasse croise à et les gaullistes à la libération pour reconstruire le pays et ça a marché et aujourd'hui pour sortir de la crise actuelle, hé bien il faut avancer plutôt dans cette direction que dans celle de la financiarisation qui nous enfonce dans la crise. Merci monsieur le président. 3000 milliards de dette. C'est la dette de la France actuellement. Ça ne tient que parce que la politique centrale européenne à des taux infiniment bas. Vraisemblablement, ce n'est pas durable pour nos systèmes ne tient que sur une politique monétaire qui est extravagante. Ce n'est pas durable. Et moi je suis comme certains d'entre vous, je conteste la méthode et je conteste aussi le moment car cette loi sur les retraites intervient à un moment où c'est ce que n'a tous lu, relu, écoutez le corps et les experts ou deux années de suite. Ce système était certes de peau mais excédentaire, personne ne l'a dit encore 2021 2022 la retraite était excédentaire. Certes, ce n'est pas durable. Certes, à terme on nous parle de déficit. on sait ce que sont que les prévisions. Par contre on sait c'est que le budget de l'État était déficitaire. De 150 milliards d'euros. Ce qu'on sait c'est que l'emprunt pour 2023 prévue pour le budget de l'État 270 milliards d'euros. Ça c'est ce sont des faits. Donc les faits, c'est que, effectivement, incapables de tenir le budget de l'État. Ben ce pouvoir propose mais bien de toucher à hein. Mais ce qui est vrai aussi c'est qu'on a le système social le plus généreux et ce système social pour qu'il évolue favorablement. Il y a besoin de la répartition, il a besoin de la capitalisation c'est comme ça que ça fonctionne ni l'un ni l'autre. Vous savez très bien que les régimes publics ont de la capitalisation. La question avant qui se pose pose c'est pas la question des retraites, avant tout, c'est la question du travail, c'est la question la création de richesses et là-dessus je ne peux pas être d'accord avec cette partie-là de l'hémicycle parce que nous sommes les plus taxés, nous sommes les plus endettés et nous sommes ce qui crée le moins de richesse mais, chers collègues. 160 milliards de déficit commercial. Est-ce que c'est un fait. Est-ce que c'est un leurre. C'est l'appauvrissement généralisé du pays que l'on traîne depuis des années et depuis 74 au budget de l'État n'a pas été

Merci monsieur le président. En fait, l'intervention du ministre qui n'a pas réellement répondu aux amendements de suppression de l'article liminaire mais il nous a quand même ouvert un Champ de réflexion assez intéressant parce que dans la même intervention. Il y a à la fois l'exaltation la valeur morale du travail et puis en même temps l'objectif clair et affirmée de ce gouvernement qui est la baisse du coût du travail. Alors le travail n'est pas une valeur morale. Monsieur le Ministre, le travail est une valeur marchande. Nécessaire, indispensable à la création de richesses et comme tout bien s'comme toute toute éléments soumis au marché il y a d'un côté celui qui veut l'acheter le moins cher possible et d'un autre côté celui qui veut le vendre le plus cher possible. Et c'est de cela dont on parle aujourd'hui parce que ce à quoi vous vous attaquez. C'est à la rémunération du travail en réalité vous n'aimez pas le travail comme vous le raconter cette cette exaltation du travail avec elle fait référence en fait vous êtes sur un terrain qui n'est pas celui de la rémunération des salariés du travail. Vous voulez qu'il soit payer le moins cher possible et en salaire puisque vous avez refusé un peu. Augmentation du SMIC que nous vous avons proposé il y a quelques mois et aussi en salaire différé parce que ce que vous appelez les charges et le coût du travail, c'est un salaire qui n'est pas versée immédiatement mais qui est déversé sous la forme de cotisations retraite pour une retraite demain ou sous la forme de cotisations d'assurance maladie pour prémunir les salariés du risque de la maladie et c'est à cela en fait que vous avez décidé avec cette réforme de vous attaquer. Mais je suis étonné d'une chose, c'est que vous êtes un homme jeune votre discours, c'est celui de Thatcher, c'est la doxa libérale que l'on entend depuis 25 ans. 25 ans. Pas une Once. Pas une Once de modernité dans votre propos, Monsieur le Ministre, la France a besoin d'autre chose que cette même rengaine sur le coût du travail et les vertus du libéralisme. Dernière explication de vote monsieur Assouline. En fait. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'il avait. Était une conviction du président de la République en 2018 2019 quand il disait que. Il fallait réformer le système des retraites. Pour répondre à aux anges sur les décennies qui viennent. Mais que le recul de l'âge était une injustice.

Il y a eu le Covid. Et il y a eu le fait que vous avez pendant 5 années et à ce moment-là en particulier. Donner beaucoup d'argent aux entreprises. On va dire. Beaucoup. Des milliards chaque année. Et ça continue. Et à un moment donné vous avez décidé et le président de la République a décidé. Hé bien d'aller chercher l'argent dans les poches des salariés et de. Rembourser quelque part ces dépenses et la dette de ces. Canaux qui ont été donnés mais parfois justifiées pour faire face à cette crise, de faire payer ceux qui étaient les premiers de corvée. Et c'est là le noeud du ce changement. Et c'est là votre réforme c'est une réforme budgétaire pour pallier à une dette, certes, mais une date relative. D'abord le fait que vous avez décidé d'épargner ce qui dans cette crise, on fait des milliards de bénéfices. Et vous êtes à côté de la plaque. À côté de ce qui est en train de se passer dans le pays parce que les gens n'arrivent plus à vivre et au lieu de répondre à ces urgences avec l'inflation et avec les salaires qui sont trop bas et les gens qui crèvent et notamment les classes moyennes vous venez leur dire conclure s'il vous plaît faire un impôt J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe communiste républicain et citoyen sur les amendements identiques de suppression. Je vous rappelle que la l'avis de la commission il est défavorable que l'avis du gouvernement, il est défavorable. Nous votons dans les conditions fixées par l'article 58 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter. Votants 344 exprimés, 344 pour 93 contre 251, le Sénat n'a pas adopté, je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise avait été 1h45 pour la suite de l'examen du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, la séance est suspendue.